La séance est reprise. Mes chers collègues, j’ai le regret de vous faire part du décès de notre ancienne collègue Brigitte Bout, qui fut sénateur du Pas de Calais de 2002 à 2011. L’ordre du jour appelle les explications de vote des groupes et le vote par scrutin public solennel sur la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir en France

que vous disposez bien de votre carte de vote et à vérifier que celle ci fonctionne correctement en l’insérant dans votre terminal de vote. En cas de difficulté, les huissiers

au premier rang desquels les collectivités locales et les fédérations du médico social. Nous désapprouvons par ailleurs le périmètre de cette proposition. Où sont les mesures pour le handicap, lequel est exclu de ce texte Pourtant, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) est bien chargée des enjeux relatifs au soutien aux personnes âgées en perte d’autonomie et aux personnes handicapées.

Cela dit, le texte transmis par l’Assemblée nationale comportait quelques avancées, certes mineures et sans cohérence d’ensemble, mais concrètes et utiles, telles que l’instauration d’un droit de visite pour les proches ou l’accès des animaux de compagnie aux Ehpad. Vous en conviendrez, la commission a supprimé une grande partie des mesures ajoutées par l’Assemblée nationale, telles que l’élaboration d’un projet d’accueil et d’accompagnement personnalisé, la remise aux personnes admises dans une structure médico sociale d’un livret d’accueil dans un format facile à lire et à comprendre, ou encore l’obligation

institutionnelle, de traiter les dérives du privé lucratif en matière d’optimisation fiscale – grâce au renforcement des contrôles –, le manque de personnel, le, la sinistralité dans le secteur des Ehpad et le virage domiciliaire.

En résumé, malgré quelques maigres mesures qui vont dans le bon sens, cette proposition de loi n’est pas satisfaisante au regard des enjeux. C’est pourquoi le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires s’abstiendra. La parole

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, depuis 2017, nous attendons impatiemment une loi sur le grand âge. Le 22 novembre 2023, la Première ministre, Élisabeth Borne, s’était engagée à présenter un projet de loi de programmation d’ici à l’été 2024. La ministre des solidarités et des familles, Aurore Bergé, qui avait annoncé un changement de méthode, a proposé d’engager une véritable coconstruction avec les parlementaires, les élus locaux et les responsables du secteur. Le 5 janvier dernier, les fédérations du secteur ont été reçues par la ministre pour échanger sur la rédaction de ce projet de loi.

avez ajouté : « Je prends l’engagement devant vous de faire une loi pour le grand âge et qu’elle soit faite et votée d’ici la fin de cette année. » Vous et vos prédécesseurs avez trop bafoué la parole publique ! Désormais, seule nous importe l’adoption d’une loi de programmation pour bâtir cette fameuse société du bien vieillir ! Nous savons Nous savons qu’une telle loi de programmation ne vous engage en rien et qu’il vous faudra trouver au moins 10 milliards d’euros pour financer l’adaptation de la société au vieillissement. Pour réaliser ces investissements, il suffit de mettre à contribution les plus hauts revenus, les revenus financiers, et les groupes qui réalisent des profits sur le dos nos aînés. Ce n’est certainement pas au travers de ce texte, qui ne prévoit que 200 millions d’euros, soit seulement 2 % des dépenses à réaliser, que nous atteindrons cet objectif. objectif. Cette proposition de loi est un coup de com’ du Gouvernement pour donner l’illusion d’avancer sur ce dossier alors qu’il n’en est rien. Pis, la majorité sénatoriale a réussi à introduire des mesures régressives dans un texte complètement creux. Cette proposition de loi, qui reprend des mesures déjà inscrites dans la convention d’objectifs et de gestion (COG) 2022 2026 entre l’État et la branche autonomie de la sécurité sociale, ne prévoit rien de novateur.

le plan Solidarité Grand Âge prévoyait que, en 2012, il y aurait huit professionnels pour dix résidents dans le budget de l’établissement. Aujourd’hui, nous en sommes toujours à six professionnels pour dix résidents Résultat, on demande aux salariés d’aller toujours plus vite, ce qui finit par épuiser le personnel. S’il y avait plus de professionnels, on réduirait les accidents du travail et on améliorerait les conditions de séjour des résidents. C’est pourquoi nous sommes convaincus de la nécessité d’augmenter les moyens en faveur de l’aide à domicile. Pour notre part, nous défendons l’objectif de recruter 200 000 personnes en Ehpad et 100 000 personnes pour le secteur de l’aide à domicile.

92 300 postes en cinq ans et d’augmenter les salaires. Vous proposez aujourd’hui d’en créer seulement 50 000 en six ans, et sans augmenter les salaires La majorité sénatoriale a supprimé la publication du taux d’encadrement dans les Ehpad au motif qu’ils rencontrent des difficultés de recrutement. Mais pourquoi les Ehpad rencontrent ils des difficultés de recrutement la pénibilité du métier, le manque de reconnaissance et un salaire moyen de 930 euros pour les aides à domicile n’attirent malheureusement pas grand monde

de leurs préconisations consistait à fixer un tarif national de l’aide à domicile à 24 euros de l’heure. Dix ans plus tard, le Gouvernement se félicite d’avoir imposé aux départements un tarif plancher à 23 euros.

pour maintenir les personnes à domicile, les familles se trouvent contraintes de chercher une place en Ehpad pour leurs proches. Elles ont deux possibilités soit elles attendent plusieurs mois dans l’espoir d’avoir une place dans un établissement public, soit elles acceptent de payer une place hors de prix dans un établissement privé. L’affaire Orpea a pourtant mis en lumière les dysfonctionnements de certains Ehpad, notamment du secteur privé lucratif, et plus largement de l’accueil des personnes âgées en situation de perte d’autonomie. En autorisant les Ehpad habilités à l’aide sociale à fixer un tarif d’hébergement différencié pour les résidents non bénéficiaires de l’aide, la majorité sénatoriale a ouvert la boîte de Pandore, et c’est extrêmement grave Désormais, les Ehpad habilités pourront moduler leurs tarifs selon les ressources des résidents et ainsi réduire davantage le nombre de places réservées aux bénéficiaires de l’aide sociale. Vous remettez en cause l’accès des familles les plus précaires à un service pourtant indispensable. En conclusion, à l’opposé du projet du Gouvernement et de la droite sénatoriale, nous défendons un véritable projet de justice sociale, visant à créer un service public de l’autonomie, financé à 100 % par la sécurité sociale, et à supprimer les exonérations de cotisations patronales. Pour l’ensemble de ces raisons, nous ne soutiendrons pas ce texte. La parole

l’horloge démographique de la France est implacable : la part des plus de 85 ans va croître de près de 90 % entre 2030 et 2050. En 2030, c’est à dire demain, la France comptera déjà 4 millions de personnes en perte d’autonomie. Ce défi, qui concernera très intimement des millions de Français et peut être chacun d’entre nous, est compliqué par la crise d’attractivité qui frappe les métiers du soin, dans un système hospitalier déjà à bout de souffle. Face à ce choc démographique, c’est d’un choc d’attractivité que nous avons besoin : sur la formation, les rémunérations des soignants, les conditions de travail et la pénibilité,

Vieillir à domicile, c’est le souhait de la très grande majorité des personnes âgées, ce que l’on peut comprendre. Ce virage domiciliaire a l’avantage d’un coût financier moindre, mais il implique une révolution celle de la politique nationale de prévention de la perte d’autonomie, domaine dans lequel nous avons des progrès à faire. En effet, 45 % des plus de 65 ans sont en bonne santé en France, contre 77 % en Suède. L’ampleur de ce défi est immense. C’est précisément pour cette raison qu’il est impératif de s’y préparer et d’engager sans tarder la loi Grand Âge, une réforme indispensable, plusieurs fois reportée. Nous restons optimistes sur sa présentation dans le courant de l’année, conformément à vos engagements, madame la ministre. En attendant, nous examinons aujourd’hui une proposition de loi de dimension plus modeste. Après un grand nettoyage de printemps en commission, nous ressortons de nos débats avec quarante articles au service de nos aînés. En réponse à la violence des situations d’isolement pendant la crise covid, le texte garantit un droit de visite quotidien dans les établissements et services sociaux ou médico sociaux (ESSMS), reprenant une initiative sénatoriale. Ces dispositions garantissent un équilibre indispensable en réservant tout de même la possibilité au directeur de l’établissement de s’opposer à une visite si elle constitue une menace pour l’ordre public ou pour la santé des résidents. Mon groupe y est favorable. Le débat qui a porté sur la présence des animaux de compagnie est loin d’être anecdotique, tant les bienfaits de la présence animale sont connus. Permettre aux établissements d’accueillir des animaux dans le cadre d’un projet d’établissement est une excellente mesure. Toutefois, excellente mesure. Toutefois, l’inscription dans la loi du droit à un animal de compagnie me semble, à titre personnel, peu réaliste au vu des contraintes. Nous saluons le financement, par la dotation soins, d’actions de prévention de la perte d’autonomie, ainsi que la généralisation de l’outil de dépistage de la perte d’autonomie (Icope). de la santé (OMS) et déjà expérimenté, il permet de repérer les facteurs de risque et de mettre en place un plan d’action, en s’adossant aux professionnels de santé et, désormais, aux nouveaux rendez vous de prévention proposés aux plus de 60 ans. C’est une excellente mesure, mais ne relâchons pas nos efforts : la prévention est un levier puissant de transformation de notre système de santé. Pour cette même raison, nous regrettons la suppression du référent prévention de l’établissement, jugé peu utile par les rapporteurs. À l’image du référent nutrition dans les Ehpad, celui ci aurait pu jouer un rôle moteur pour déclencher des actions de prévention dans les établissements. Nous regrettons également que notre amendement prévoyant le remboursement de l’activité physique adaptée pour les personnes en perte d’autonomie ait été déclaré irrecevable. Nous avons récemment voté, grâce au soutien du Gouvernement, la prise en charge par l’assurance maladie de l’APA pour les patients atteints de cancer. Pourquoi ne pas envisager la même mesure pour les personnes âgées, en prévention de la perte d’autonomie ? Madame la ministre, profitons de cette année olympique où le sport a été décrété grande cause nationale pour nous engager sur la question du sport santé et de l’activité physique adaptée au service des plus fragiles. Ce texte contient par ailleurs des mesures intéressantes pour prévenir la maltraitance des personnes vulnérables, des maltraitances organisées, comme le scandale Orpea nous en a révélé, mais aussi des maltraitances plus institutionnelles, par manque de soignants, de formation, ou encore par épuisement professionnel. Ainsi, nous saluons la création d’une cellule départementale de recueil et de suivi des signalements, ainsi que l’élargissement de la Conférence nationale de santé (CNS) à la question de la maltraitance. J’en viens maintenant à l’organisation territoriale de l’offre. Un service public départemental de l’autonomie (SPDA) sera créé pour mieux orienter les personnes, faciliter leurs démarches et coordonner les services. Nous insistons sur l’importance de laisser de la souplesse à cet outil pour mieux l’adapter aux réalités locales. La version adoptée convient à notre groupe, avec un plan trisannuel et la possibilité de définir des territoires de l’autonomie à l’échelon infradépartemental. Au risque de me répéter, la décentralisation en matière de santé est un chantier indispensable et urgent à mener, tant les besoins et les réalités varient d’un bassin de vie à l’autre. Je conclus sur le nerf de la guerre, l’attractivité des métiers. Si les revalorisations salariales ne peuvent figurer dans une proposition de loi, quelques mesures intéressantes sont à saluer. Je pense notamment à l’expérimentation de la tarification forfaitaire des services autonomie à domicile (SAD). Conformément à notre amendement et au souhait des départements, cette expérimentation débutera en 2025 et pour deux ans, avant une possible généralisation. La question de la mobilité n’est pas oubliée, et c’est heureux. Une aide annuelle sera versée par l’État aux départements qui soutiennent les aides à domicile dans l’obtention du permis de conduire, dans leurs déplacements, mais aussi dans des temps collectifs d’échanges entre professionnels, ainsi que l’attendait la profession. Ces 100 millions d’euros amélioreront le quotidien des professionnels – qui le méritent, tant leur présence auprès de nos aînés est essentielle. Enfin, je n’insisterai pas sur la nouvelle carte pour les intervenants à domicile. Elle était attendue, mais elle revêt un caractère essentiellement symbolique et ne répondra pas aux besoins du secteur, à moins qu’un décret ne vienne effectivement l’assortir d’avantages concrets, notamment en matière de mobilité. En conclusion, si elle n’est pas la grande loi attendue pour adapter notre société aux immenses défis du vieillissement, cette proposition de loi contient de bonnes idées auxquelles le groupe RDSE apportera sa voix.

alors que nous arrivons à la fin de l’examen du texte sur le bien vieillir en France, le groupe RDPI se satisfait que nos discussions aient été l’occasion de débats de qualité et qu’elles aient pu redonner à cette proposition de loi une forme plus intelligible en réduisant le nombre de ses articles. Nous nous réjouissons des diverses avancées obtenues, notamment pour les aides à domicile, avec la carte professionnelle ou encore les aides à la mobilité. Nous sommes également satisfaits de l’adoption de différents amendements du groupe RDPI, qui ont enrichi le texte, que ce soit sur le service public départemental de l’autonomie ou encore sur la prise en compte des spécificités des territoires ultramarins dans les aides à la mobilité. Néanmoins, nous regrettons que les rapporteurs n’aient pas entendu nos arguments sur plusieurs sujets, notamment sur le rétablissement des dispositions relatives au pouvoir du juge des tutelles de nommer un tuteur ou un curateur de remplacement pour les personnes âgées, ou encore sur le statut des Ehpad. Nous espérons que la commission mixte paritaire trouvera un accord sur ces questions. Madame la ministre, nous aurions aussi aimé avoir des chiffres plus précis sur le financement de cette proposition de loi. Je souhaite également évoquer le sujet de l’outre mer. Lors de la discussion générale, madame la ministre, vous m’aviez répondu que vous vous engagiez à agir avec ambition pour répondre aux enjeux plus spécifiques du vieillissement en outre mer.

touchant à la fois à la coordination nationale des politiques publiques, à une lutte plus efficace contre la maltraitance, ainsi qu’à un meilleur accompagnement des professionnels du secteur. Nous voterons donc sans hésitation ce texte. Madame la ministre, nous attendons néanmoins que la promesse du Gouvernement de présenter une loi sur le grand âge d’ici à la fin de l’année se concrétise, et nous serons alors des partenaires exigeants sur le sujet.

continuer d’agir sur le financement des politiques publiques sur le grand âge. Il nous faut en effet trouver 10 milliards d’euros par an d’ici à 2030, malgré les financements toujours plus importants que le Gouvernement a consacrés à la branche de la sécurité sociale dédiée à l’autonomie créée en 2020 – en témoigne encore l’affectation de 0,15 point de contribution sociale généralisée (CSG) à son financement, soit 2,4 milliards d’euros supplémentaires par an, pour atteindre 42 milliards d’euros de dépenses en 2026. Nous devons également redonner de l’attractivité au secteur, qui en manque cruellement depuis des années, et, enfin, rester vigilants sur le contrôle des Ehpad pour que les scandales récents ne se reproduisent plus.

le groupe sénatorial de la majorité présidentielle est volontariste pour avancer sur le sujet du grand âge. Vous pouvez donc compter sur nous pour être à vos côtés, madame la ministre. Nous devons continuer de montrer à nos aînés ainsi qu’à celles et ceux qui les soutiennent que nous nous occupons d’eux au quotidien et que nous pouvons œuvrer ensemble en faveur de leurs droits. Comme le disait Montaigne, « la vieillesse n’est pas une maladie, mais le plus grand des mérites ». La parole

nous l’avons dit la semaine dernière : certaines dispositions de la proposition de loi portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir en France, prises isolément, vont plutôt dans le bon sens. Il manque cependant une vision globale, celle qu’aurait dû contenir la grande loi annoncée depuis six ans par le Président Macron, texte que nous attendons toujours. Ce texte aborde le sujet essentiel du vieillissement et nous questionne sur la capacité de notre société à y faire face. Il est plus qu’urgent de répondre à la peur de celles et de ceux qui vieillissent, qui craignent de se trouver isolés et de ne pas avoir les moyens d’affronter la perte d’autonomie. Nous sommes face à un défi majeur, auquel notre société doit répondre – et ce n’est évidemment pas cette proposition de loi qui permettra de le faire… Conscients des légitimes attentes de nos concitoyens, les sénateurs du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ont formulé de nombreuses propositions constructives, par voie d’amendement, qui n’ont pas trouvé d’écho favorable. Nous le regrettons. Surtout, les débats en séance ont permis de mettre en lumière certains points de vigilance. C’est le cas de l’article 1 F, qui crée une obligation pour les Ehpad publics autonomes de coopérer dans le cadre d’un nouveau type de groupement, à savoir les groupements territoriaux sociaux et médico sociaux Si nous sommes tous convaincus de la nécessité que les établissements coopèrent au service des personnes à accompagner, il ne faudrait pas que la création de cette obligation aboutisse à la même situation que celle qui a suivi la mise en place des groupements hospitaliers de territoire Plus largement, c’est une évidence : avant de réfléchir à l’organisation territoriale, aux regroupements possibles et de fixer des obligations s’imposant à tous, il eût été préférable que notre pays se fixe un cap, une stratégie en matière d’autonomie et d’accompagnement des personnes âgées, et que nous évoquions le financement. Se réunir pour échanger, c’est bien, surtout s’il y a un projet réfléchi qui part du territoire ; cependant, sans moyens, nous risquons de ne pas aller très loin. De même, nous regrettons la suppression de toute une série d’articles comme le 11 B, qui prévoyait de déroger au renouvellement par tacite reconduction de l’autorisation d’un ESSMS sur la recommandation de l’évaluation externe ou si le contrôle réalisé par une des autorités compétentes le mentionne dans ses conclusions. À la suite de la publication du livre, de Victor Castanet, l’ensemble de la société française et ses responsables politiques ont été scandalisés par l’insuffisance des contrôles des Ehpad, notamment des établissements à statut privé à but lucratif. Or une minorité d’entre eux voient leur autorisation d’ouverture tacitement reconduite depuis des années, malgré les alertes des financeurs – agences régionales de santé et départements – lors des contrôles. Nous voulions que ce ne soit plus possible. Nous aurions tout autant souhaité rétablir l’article 11 D, qui instaurait une mesure de régulation économique garantissant que les bénéfices réalisés par les Ehpad privés lucratifs soient en partie sanctuarisés et fléchés pour participer à l’amélioration de la qualité de l’hébergement des personnes âgées. l’article 11 , qui permettait d’automatiser le régime des sanctions à l’encontre des établissements qui ne respecteraient pas leurs obligations de qualité de soins et d’accompagnement à la suite des injonctions qui leur seraient adressées par les autorités compétentes. Nous souhaitions enfin rétablir l’article 12 , en vue d’obliger les Ehpad privés et leurs gestionnaires à s’inscrire dans le cadre du statut de la société à mission, et ainsi renforcer les exigences de ces structures privées en matière d’engagements d’intérêt général et d’utilité sociale. Le rétablissement de ces articles a malheureusement été rejeté par la majorité sénatoriale. Certes, certaines mesures vont plutôt dans le bon sens, comme la création d’un service public départemental de l’autonomie et d’une carte professionnelle pour l’ensemble des intervenants au domicile des personnes âgées handicapées, sous condition, quel que soit leur statut. Nous avançons également sur la prise en charge des frais de mobilité des professionnels, surtout après l’engagement pris de soutenir la branche de l’aide à domicile dans la revalorisation de son barème kilométrique, la création d’un fonds de soutien à la mobilité des aides à domicile doté de 100 millions d’euros par an. Toutefois, là encore, cela ne peut pas suffire. Les tensions existantes en matière de ressources humaines dans le secteur médico social sont autant causées par le bouleversement du rapport au travail touchant l’ensemble de la société que par de lourdes difficultés structurelles : manque de reconnaissance, droit social inadapté, risques professionnels élevés, etc. À ces dernières, le texte n’apporte pas de réelles réponses,

bien conscients que tout ce qui avait été promis à la représentation nationale il y a encore quelques semaines ne tient plus. Ainsi, nous nous interrogeons sur le respect de l’engagement relatif au vote d’une loi de programmation pluriannuelle pour le grand âge avant la fin de l’année 2024. Nous aurions aimé vous entendre, madame la ministre, reprendre cet engagement à votre compte de façon claire et ferme. Que de temps perdu, alors qu’il y a urgence à agir, investir, former, innover !

Vouloir « bâtir une société du bien vieillir » suppose de proposer une prise en charge adaptée qualitativement et financièrement aux besoins des personnes vieillissantes. Force est de constater que la proposition de loi adoptée par nos collègues députés constitue davantage un catalogue de mesures diverses qu’une véritable réforme des politiques de soutien à l’autonomie. Nous avons abordé l’examen de ce texte au pas de course avec la volonté de le recentrer sur son contenu utile en faveur des personnes âgées ou en situation de handicap. Pour ce faire, nous avons supprimé une trentaine d’articles et mis en évidence des mesures structurantes. Permettez moi de revenir sur les points qui nous semblent importants. En matière de gouvernance et de pilotage, nous avons supprimé la nouvelle conférence nationale de l’autonomie, considérée comme redondante. En revanche, nous avons approuvé la création du service public départemental de l’autonomie. Certes, le SPDA ne va pas bouleverser la gouvernance territoriale des politiques de l’autonomie, mais le texte permet de rendre ce dispositif souple et facilement adaptable aux spécificités de chaque territoire. En outre, le maintien à domicile est inscrit comme l’un des objectifs du SPDA, au même titre que le suivi dans la durée des personnes en situation de dépendance. En matière de prévention de la perte d’autonomie, la généralisation du programme Icope constitue une avancée.

Par ailleurs, conscients de l’importance des animaux de compagnie dans le quotidien des personnes en perte d’autonomie, et au déchirement que peut représenter l’admission dans un Ehpad, nous avons fait en sorte de concilier l’accueil des animaux domestiques des résidents avec les contraintes propres aux établissements. S’agissant du signalement des cas de maltraitance, nous avons prévu la création d’une cellule sous l’autorité conjointe du conseil départemental et de l’agence régionale de santé. Cette cellule inclura également les centres Allo Maltraitance (Alma), déjà dotés d’un savoir faire dans le recueil et l’évaluation des situations de maltraitance, notamment au moyen du numéro 3977. Le soutien au virage domiciliaire passe par l’amélioration de l’attractivité du métier d’aide à domicile. Nous regrettons la faible portée des mesures. Nous avons décidé de soutenir la mobilité des personnels du secteur en rendant éligibles aux aides de la CNSA les actions des départements en faveur du financement du permis de conduire. Malgré les améliorations adoptées par notre assemblée, cette proposition de loi ne répond que très partiellement aux enjeux du vieillissement de la population. Les réponses sont en effet encore trop timides, notamment en matière de prévention de la perte d’autonomie de la personne âgée, de la personne handicapée et des proches aidants. Il en est de même pour la question du virage domiciliaire, pourtant appelé de leurs vœux par 90 % de nos concitoyens.

La prévention de la perte d’autonomie est un volet central. Il est primordial de généraliser au plus tôt la mise en place de l’Icope pour repérer les facteurs de risque et prévoir un plan d’action personnalisé avec les professionnels de santé.

enfin, vers les unités de soins de longue durée (USLD). Il s’agirait ainsi de préparer cette transition en gardant un cap. Certes, les moyens sont nécessaires et attendus par tous ; mais pour mettre en œuvre ces propositions, il nous faut des professionnels formés, compétents, reconnus, rémunérés et un taux d’encadrement adéquat. L’attractivité des métiers y contribuera fortement. Concernant les aides à domicile, formation, statut, rémunération et mobilité sont les mots clés pour permettre l’amélioration de la prise en charge domiciliaire.

nécessaire de renforcer la formation. Les 50 000 postes que vous voulez créer dans les Ehpad et les services d’aide et d’accompagnement à domicile ne verront pas le jour en quelques mois seulement. Il faut peut être aussi penser à valoriser le métier d’aide soignant à domicile. Enfin, la qualité de prise en charge de la personne âgée et de la personne handicapée et la reconnaissance des proches aidants ne pourront s’améliorer qu’avec le concours de tous les professionnels – c’est à dire les soignants et les travailleurs sociaux –, des usagers et de leur famille, et, bien sûr, des collectivités locales et des élus. Sur toutes les travées de notre assemblée, nous sommes convaincus que l’autonomie et le grand âge sont des enjeux centraux pour l’avenir de notre société. Nous attendons donc avec impatience, depuis six ans maintenant, une loi pour répondre aux différents défis du vieillissement. Pour conclure, le groupe Les Républicains votera ce texte dans sa version modifiée par le Sénat. La parole

garantir le consentement libre et éclairé de nos aînés, pour qu’ils puissent vivre. La société du bien vieillir que nous voulons sera fondée sur l’accompagnement à domicile avec des aménagements financés pour que le logement soit adapté aux besoins de nos aînés. Il faudra développer et améliorer la mise en réseau de tous les acteurs de ce processus. Nous devons aussi penser l’Ehpad de demain et écouter les demandes du secteur, mais aussi des familles et des personnes âgées elles mêmes.

Que dire sur la vision du Gouvernement de l’Ehpad de demain ? En effet, l’Ehpad doit changer et être repensé pour mieux individualiser l’accompagnement et la volonté de chaque résident, à l’heure où beaucoup d’établissements sont obligés de standardiser les parcours de soins, faute de moyens, de personnel, mais aussi d’ambition politique, madame la ministre.

Madame la présidente,

le nombre de personnes de plus de 85 ans va doubler entre 2020 et 2040. D’ici à 2050, on comptera même, selon les estimations, plus de 4,8 millions de personnes âgées de plus de 85 ans. Le nombre de personnes dépendantes approchera quant à lui les 2 millions d’ici à 2040. Il est un chiffre que l’on cite moins, et qui est peut être, pourtant, au moins aussi parlant : on compte trente fois plus de centenaires aujourd’hui dans notre pays que dans les années 1970. Il n’y a donc pas besoin d’être fin analyste pour comprendre à quel point notre pays vieillit, et que le vieillissement n’est pas le défi de demain, mais, d’ores et déjà, d’ores et déjà, celui d’aujourd’hui. C’est donc d’un projet de loi d’ampleur, à la hauteur des enjeux et avec les moyens corrélatifs, que les Français ont besoin. Nous, parlementaires, l’attendons. Adaptation des logements, des établissements médico sociaux et de l’urbanisme, aide à la mobilité, formation du personnel soignant, prise en compte des disparités importantes selon les territoires – je pense notamment aux outre mer : les enjeux d’adaptation au vieillissement sont nombreux. La proposition de loi que nous devons voter aujourd’hui est elle ce texte tant attendu ? Malheureusement, non. Elle dresse les contours de quelques améliorations nécessaires, mais sans aller assez loin. Surtout, elle ne donne aucune perspective financière. Le titre de cette proposition de loi a d’ailleurs été revu en commission, pour l’adapter très justement à un contenu bien moins ambitieux que ce qu’elle affichait initialement. Arrivé au Sénat avec soixante cinq articles, le texte pouvait laisser espérer des avancées majeures. En réalité, il contenait beaucoup d’articles inutiles, symboliques, de portée réglementaire ou même déjà satisfaits par le droit en vigueur. Le travail effectué en commission a permis de ramener cette proposition de loi au rang d’un texte législatif. Cela dit, on comprend bien que la longueur et le contenu du texte transmis au Sénat n’étaient que le reflet de l’émotion suscitée par le scandale qui a éclaté au sein des Ehpad en 2022, faisant lui même suite au traumatisme encore récent des restrictions lors de la crise sanitaire. angoisse légitime a été suscitée par les récits les plus durs que l’on puisse imaginer. Ceux ci nous renvoient inévitablement à la peur de la dépendance, celle de nos proches,

nous avons rappelé, avec le travail effectué dans notre Chambre haute, que le rôle du Parlement n’est pas de légiférer sous le coup de l’émotion, mais de garder la tête froide pour prendre des décisions raisonnées et raisonnables.

Je souhaite donc remercier tous ces professionnels qui, chaque jour, parfois au prix de leur propre santé, font la différence auprès de nos aînés en leur apportant gentillesse et bienveillance. J’ai une pensée toute particulière pour les salariés et bénévoles du Village Santé Saint Joseph, dans les Mauges. Ce texte, s’il ne propose pas de bouleversements majeurs, offre néanmoins quelques avancées. La création d’un service public départemental de l’autonomie est une mesure de bon sens qui permettra un pilotage cohérent de la prise en charge de la perte d’autonomie à l’échelle du département. Il permettra d’orienter les personnes âgées, les personnes en situation de handicap et leurs proches, en s’assurant du bon suivi des dossiers par les services compétents. Nous formons le vœu qu’il contribue ainsi, par une meilleure coordination des acteurs, à faciliter ce qui peut parfois ressembler à un parcours du combattant pour les usagers. J’aurais préféré, pour ma part, que l’instauration d’une conférence nationale de l’autonomie soit maintenue, car celle ci aurait placé ce thème au centre des préoccupations de plusieurs ministères, garantissant ainsi sa prise en compte. Dès l’année prochaine, les départements volontaires auront la possibilité d’expérimenter le financement des services autonomie à domicile par des dotations forfaitaires, au lieu de facturations à l’heure.

Cette carte reste néanmoins symbolique : la meilleure reconnaissance de ces professions passe avant tout par une revalorisation de leurs rémunérations. Sur ce point, l’aide financière accordée aux départements pour aider à la mobilité des intervenants à domicile va dans le bon sens, et nous nous félicitons que le permis de conduire y ait été intégré. Nous saluons aussi l’adoption d’un amendement de notre collègue Pierre Jean Rochette, qui a permis la suppression d’un article ajoutant des contraintes administratives aux Ehpad, sans rendre plus efficace la lutte contre la maltraitance. Vous l’avez compris, notre groupe votera en faveur de ce texte ; pour autant, madame la ministre, nous attendons de pied ferme un projet de loi pour le grand âge contenant une projection précise pour les années à venir et apportant des moyens chiffrés.

Je tiens à remercier l’équipe du Sénat ainsi que celle du cabinet ministériel, qui ont su travailler en bonne intelligence sur des sujets parfois sensibles et dans un contexte de remaniement ministériel assez singulier. Je remercie aussi mon collègue Jean Sol, avec qui j’ai eu l’honneur de travailler. Cela nous a permis d’avancer sur le texte de Mme Aurore Bergé, initialement intitulé « proposition de loi portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir ». Il s’agit d’une préoccupation majeure des Français. Ce texte, initialement composé de quatorze articles, en comptait soixante cinq à l’issue de son examen par l’Assemblée nationale. Notre objectif a été de le recentrer sur les dispositifs véritablement utiles pour répondre aux enjeux liés au vieillissement de la population et à l’accompagnement des personnes en situation de handicap. C’est pourquoi nous avons supprimé plusieurs articles dont les dispositions étaient déjà satisfaites ou relevaient du pouvoir réglementaire. Revenons sur les enjeux auxquels je m’intéresse particulièrement renforcer le droit au respect de la vie privée et familiale, améliorer la lutte contre la maltraitance et garantir des conditions d’hébergement et d’habitat ainsi que des prestations de qualité dans l’aide à domicile grâce à des professionnels accompagnés et soutenus dans leurs pratiques. Je salue la reconnaissance d’un droit de visite dans les Ehpad, les ESSMS ou encore les établissements de santé. La commission a ainsi introduit dans le texte les dispositions de la proposition de loi du président Bruno Retailleau Nous avons par ailleurs supprimé l’article 3 A, lequel consacrait, dans un dispositif inopérant, le droit à une vie affective et sexuelle pour les usagers des établissements médico sociaux. sociaux. Celui ci est déjà garanti par le droit en vigueur et cet article ne nous semble pas adapté au respect de l’intimité des résidents ; il ne répond pas, en outre, aux difficultés pouvant être rencontrées en structure médico sociale : séparation d’avec le conjoint, assurance du consentement en présence de troubles psychiques de la personne, etc. Je suis néanmoins satisfaite que son examen mette en lumière ce sujet encore largement tabou. L’article 4 prévoit la création d’une cellule départementale de recueil et de suivi des signalements de maltraitance envers les personnes majeures vulnérables du fait de leur âge ou de leur handicap. Placées sous l’autorité conjointe du président du conseil départemental et de l’ARS, ces cellules visent à centraliser les signalements adressés au numéro d’alerte national 3977, créé en 2008.

En revanche, nous ne sommes pas favorables à imposer à tous les Ehpad la création d’un comité d’éthique, puisque cela introduirait une organisation trop lourde et, dans certains cas, Pour accueillir les personnes en toute sécurité au sein des structures médico sociales, le contrôle des antécédents judiciaires des intervenants, bénévoles et professionnels, a été renforcé une première fois par la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants. Je me réjouis que le Sénat ait adopté, à l’article 5 A, de nouvelles dispositions sécurisant le criblage de ces antécédents. Il sera ainsi possible de suspendre temporairement une personne condamnée non définitivement ou mise en examen.

sous peine de suspension automatique de ses activités. Toutefois, la procédure entourant la suspension temporaire des personnes condamnées non définitivement ou mises en examen d’une telle mesure, il était plus sage de ne pas adopter dans la précipitation un tel dispositif et de travailler, dans la suite de la navette, à une rédaction mieux adaptée. En ce qui concerne le secteur du domicile, j’approuve la création d’une carte professionnelle pour les intervenants à domicile, une mesure cependant essentiellement symbolique. La majorité de ces professionnels ne disposant d’aucun titre ou diplôme, la commission a prévu, à juste titre, d’en ouvrir le bénéfice aux personnes justifiant obligatoirement de deux années d’exercice professionnel. Les facilités offertes par cette carte devront toutefois être précisées par un décret. décret. Je suis heureuse de l’adoption de mon amendement visant à aider les professionnels intervenant à domicile à obtenir le permis de conduire, une disposition indispensable pour les habitants des communes rurales, dans lesquelles les contraintes de mobilité constituent un véritable obstacle au recrutement. Le regroupement des catégories existantes de services à domicile en une unique catégorie dénommée SAD, que nous avons voté dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, implique une transformation qui se révèle difficile en pratique pour les services, notamment pour Ces derniers disposant d’un délai de deux ans pour fusionner ou se regrouper avec un SAD existant, ils craignent de disparaître s’ils ne parviennent pas à obtenir à temps une autorisation. L’article 8 vise à répondre à ces inquiétudes en permettant aux Ssiad de conventionner avec un SAD pendant une durée de trois ans, sans demander de nouvelle autorisation. Il prévoit en outre un délai supplémentaire pour les Ssiad recevant un refus d’autorisation, que nous avons proposé d’étendre à deux ans. chers collègues, vous avez relayé les doutes de vos territoires à l’égard de ce processus en votant en faveur d’un assouplissement du cadre des services autonomie à domicile. Je partage votre préoccupation. Pour autant, il ne semble pas opportun de remettre en cause cette réforme, déjà bien engagée. Nous veillerons, dans la suite de la navette, à garantir un meilleur accompagnement des Ssiad dans la gestion de cette période transitoire. L’article 13 A tend à garantir la qualification des locaux dans lesquels sont constitués les habitats inclusifs en bâtiment d’habitation pour l’application de la réglementation en matière de sécurité contre les risques d’incendie. Cela permettra de leur épargner les contraintes liées au risque de requalification en établissement recevant du public, qui pourrait menacer le financement de l’habitat inclusif Dans le but de soutenir le développement de ce type d’habitat, je suis favorable au renforcement de la sécurité juridique ; pour autant, ce sujet me semble mériter une réflexion plus approfondie dans les années à venir. Pour terminer, nous attendons impatiemment le projet de loi de programmation pluriannuelle pour le grand âge et nous veillerons à ce que celui ci soit à la hauteur des attentes de l’ensemble des acteurs du soutien à l’autonomie. Ce texte ne devra pas faire l’impasse sur la gouvernance non plus que, surtout, sur la répartition des moyens financiers. Il est indispensable de préciser qui va payer quoi, afin d’assurer une coordination sereine entre les différentes instances : ARS, départements et CNSA.

vous est donné de cette mise au point, mon cher collègue. Elle figurera dans l’analyse politique du scrutin concerné. L’ordre du jour appelle la discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi, modifiée par l’Assemblée nationale, visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales

l’enfance a été placée par le Président de la République au nombre de nos priorités et la protection des droits de l’enfant est au cœur de la feuille de route du Gouvernement, qui en a fait un engagement prioritaire. C’est la raison pour laquelle je me réjouis que la proposition de loi visant à mieux protéger les enfants victimes de violences intrafamiliales soit discutée en deuxième lecture aujourd’hui par la Haute Assemblée.

lequel modifie l’article 378 2 du code civil afin d’étendre le mécanisme de suspension de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi ou condamné.

au cas de la poursuite ou de la condamnation d’un parent pour crime commis sur la personne de l’autre parent ou pour agression sexuelle incestueuse ou crime commis sur la personne de l’enfant. Cette rédaction ne manque pas d’intérêt et je veux ici saluer chaleureusement le travail de la rapporteure, Mme Marie Mercier. Tout d’abord, il aurait été impensable d’introduire une hiérarchie entre les crimes dont un enfant peut être victime et de prévoir la suspension de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite pour certains d’entre ceux ci et non pour d’autres. Nous pouvons nous féliciter que la nécessité de viser tous les crimes commis sur l’enfant ait été entendue lors des débats parlementaires et de nouveau par la commission des lois du Sénat. Inversement, il me semble qu’il aurait été tout aussi inopportun de viser n’importe quel délit. La suspension automatique de l’exercice de l’autorité parentale dès le stade des poursuites, et alors que le parent est présumé innocent, doit être réservée aux infractions les plus graves. Il y va de la constitutionnalité et de la conventionnalité du dispositif. Il est donc cohérent de limiter celui ci aux agressions sexuelles incestueuses. À cet égard, il me semble tout à fait utile, dès lors que la simple décision de poursuivre permet de déclencher ce mécanisme, de préciser que les actes de poursuite émanent du procureur de la République ou du juge d’instruction. Une telle règle procédurale permet de prévenir les constitutions de partie civile ou les citations directes abusives par l’autre parent. Ces éléments, fondamentaux pour l’équilibre du dispositif, font d’ailleurs consensus entre les deux assemblées, ce dont je me réjouis. En revanche, la rédaction votée par votre commission a maintenu le caractère provisoire du mécanisme de suspension automatique de l’exercice de l’autorité parentale. Elle prévoit que cette suspension opère jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales (JAF) et pour une durée maximale de six mois. Il y a là un premier point de débat entre les deux chambres, l’Assemblée nationale ayant souhaité que la suspension se poursuive non pas pour une durée maximale de six mois, mais jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, familiales, le cas échéant saisi par la personne poursuivie, jusqu’à la décision de non lieu du juge d’instruction, ou encore jusqu’à la décision ou l’arrêt pénal. Ces deux approches traduisent la recherche d’équilibre entre les droits du parent et la protection des enfants. Des amendements posent ce débat, avec des rédactions préservant, à mon sens, la protection maximale de l’enfant, dans la mesure où nous entendons laisser aux parents la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales. Par ailleurs, votre commission a supprimé l’alinéa 2 de l’article 1, lequel vise à créer un dispositif de suspension automatique de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement du parent condamné pour violence conjugale ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) de plus de huit jours, lorsque les faits se sont déroulés en présence de l’enfant. Ce dispositif étant réservé aux faits les plus graves commis en présence de l’enfant, nous avions atteint, à mon sens, un équilibre proportionné pour conserver un maximum de garanties aux bénéfices de ce dernier. Telles sont finalement les deux seules dispositions qui ne recueillent pas, à cette heure, l’accord de vos deux assemblées et qui seront évidemment au cœur de nos débats cet après midi. L’article 2 fait désormais consensus, dans une rédaction qui constitue, à n’en pas douter, une avancée indéniable en matière de protection des enfants, puisque le juge pénal aura l’obligation – et non plus la simple faculté, comme cela est actuellement le cas – de retirer l’autorité parentale ou son exercice, en cas de condamnation du parent pour les infractions les plus graves commises sur son enfant ou sur l’autre parent. L’article 2, qui semble lui aussi faire consensus, puisque votre commission ne l’a pas modifié, prévoit que le parent privé de l’exercice de l’autorité parentale et de ses droits de visite et d’hébergement à la suite d’une condamnation pénale ne pourra pas saisir le juge aux affaires familiales afin de se voir restituer cet exercice et ses droits de visite et d’hébergement avant l’expiration d’un délai de six mois. Cet article est conforme à l’esprit de cette proposition de loi : renforcer la protection de l’enfant. Enfin, l’article 3, qui fait lui aussi consensus, a pour objectif simple simplifier le code pénal, par l’introduction d’un article unique regroupant toutes les dispositions applicables en matière de retrait de l’autorité parentale d’un contenu identique aux dispositions figurant dans le code civil. Tel est donc le texte qui vous est présenté aujourd’hui, Au delà des quelques divergences qui demeurent entre les deux chambres, ce texte n’en doutons pas est très attendu par nos concitoyens, parce qu’il renforce la protection des plus vulnérables d’entre nous, parce qu’il est de notre devoir de protéger l’enfant victime de son parent agresseur, et, enfin, parce que le foyer doit toujours rester un lieu où l’enfant peut grandir en paix et en sécurité.

La commission des lois vous propose d’en adopter quatre supplémentaires afin de concentrer les débats sur l’article 1, qui pose l’importante question de l’intervention du juge pour apprécier l’intérêt de l’enfant. L’article 2 de la proposition de loi tend à modifier l’article 378 du code civil pour rendre plus automatique, mais sans l’imposer au juge – ce qui est important le retrait de l’autorité parentale ou de l’exercice de l’autorité parentale en cas de condamnation pour crime ou agression sexuelle incestueuse sur l’enfant ou pour crime sur l’autre parent.

La commission a accepté cette formulation, dans la mesure où les juridictions conserveraient malgré tout le choix de moduler leurs décisions en fonction de l’intérêt de l’enfant, apprécié, à charge pour elles de le motiver spécialement. qui concerne l’article 3, les députés ont repris notre idée de rassembler en un seul article du code pénal l’ensemble des dispositions relatives au retrait de l’autorité parentale par les juridictions pénales, ce qui devrait en faciliter l’application. Ils ont choisi d’en faire une disposition miroir de l’article 378 du code civil sans procéder par renvoi, ce qui ne semble pas nuire à l’intelligibilité et à l’effectivité recherchées.

viens à présent à l’article 1 de la proposition de loi, que les députés ont adopté dans les mêmes termes que leur texte de première lecture. Cet article modifie l’article 378 2 du code civil pour élargir les cas de suspension de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement aux cas de crime ou d’agression sexuelle incestueuse commis sur l’enfant, tout en modifiant le régime. C’est sur ce dernier point que nous avons un désaccord. effet proposé que, en cas de poursuites, de mise en examen ou de condamnation pour un crime commis sur l’autre parent ou de crime ou agression sexuelle incestueuse commis sur l’enfant, l’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement soient suspendus

Les députés ont également prévu un régime spécifique en cas de condamnation pour des violences volontaires sur l’autre parent ayant entraîné une ITT de plus de huit jours, lorsque l’enfant a assisté aux faits. Comme en première lecture, nous avons accepté d’étendre le mécanisme de suspension provisoire avant tout jugement au cas de crime ou d’agression sexuelle incestueuse commis sur l’enfant.

Nous avons toutefois souhaité maintenir le caractère provisoire de la suspension dans les conditions actuelles, c’est à dire pour une durée maximale de six mois, jusqu’à la décision du JAF, qui doit être saisi par le procureur de la République dans les huit jours.

enfin écarté le dispositif spécifique proposé en cas de condamnation pour violences volontaires ayant entraîné une ITT de plus de huit jours, lorsque l’enfant a assisté au fait. Les juridictions doivent déjà se prononcer sur l’autorité parentale en cas de condamnation au titre de cette infraction, les enfants témoins étant des covictimes, ainsi que les désigne l’intitulé de la proposition de loi. Mes chers collègues, c’est bien sur une question d’équilibre que nous aurons à nous prononcer lors de l’examen des différents amendements qui nous sont soumis. Contrairement

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, nous discutons aujourd’hui d’une proposition de loi nécessaire, dont l’ancien président de la Ciivise, Édouard Durand, disait qu’elle était à la fois conforme aux principes et à la raison. Les chiffres sont édifiants, et nous ne pouvons pas dire que nous ne les connaissons pas : 400 000 enfants vivent dans un foyer où s’exercent des violences intrafamiliales de manière permanente 60 000 enfants sont victimes de violences sexuelles. Dans mon département, La Réunion, chaque jour, sept enfants sont identifiés comme étant en danger par la cellule de recueil des informations préoccupantes, et les signalements directs ont augmenté de 60 % depuis 2019. Cette proposition de loi comble un vide juridique en matière d’autorité parentale des parents coupables de violences criminelles. Parce que la saisine du juge aux affaires familiales n’est pas toujours effective, parce que les délais pour obtenir une date d’audience du juge aux affaires familiales sont trop longs, le retrait et la suspension de l’autorité parentale restent aujourd’hui des possibilités trop peu appliquées. Il est donc urgent de rappeler dans la loi que tout enfant doit être protégé, y compris de ses parents quand il le faut. La certitude selon laquelle le lien entre l’enfant et son parent doit être maintenu à tout prix irrigue encore trop souvent la pensée des magistrats. Oui, cette certitude doit être remise en question. Non, un parent qui viole son enfant ne peut pas continuer à avoir l’autorité parentale sur lui. L’intérêt supérieur de l’enfant doit l’emporter sur le droit des parents d’influer sur la vie de cet enfant. L’intérêt supérieur de l’enfant et sa protection doivent nous guider, C’est ce que nous enseignent les très nombreux témoignages recueillis par la Ciivise, notamment de mères s’inquiétant de laisser leur enfant repartir chez le père incestueux. Un enfant obligé d’aller chez le parent violent en attendant le jugement continuera d’y subir violences, emprise, influences et menaces. Il cessera alors d’un coup d’en parler. La suspension de l’autorité parentale n’est pas seulement nécessaire à la libération de la parole : elle l’est aussi pour protéger les enfants. Plus qu’écouter, il faut protéger des conséquences dramatiques qu’ont les violences sur le développement, sur la construction et la scolarité des enfants. On sait ce qu’engendrent les violences en termes de chocs traumatiques, de phénomènes de dissociation, de troubles de la mémoire et de conduites à risque. On sait que l’exposition précoce à ces violences constitue le premier facteur de risque de suicide, de dépression, de précarité et qu’elle accroît le risque de subir de nouvelles violences ou d’en faire subir à son tour. à son tour. Une étude de l’ONU montre qu’une femme qui a subi des violences physiques et sexuelles dans l’enfance a dix neuf fois plus de risques de subir des violences conjugales ou sexuelles à l’âge adulte par rapport à une femme qui n’en a pas connu homme qui a connu le même type de violences a quatorze fois plus de risques d’en commettre à son tour. En définitive, tout plaide pour une mise en sécurité rapide et automatique des enfants victimes, pour une prise en charge plus précoce afin de limiter les conséquences sur la santé des victimes. Nous devons garder en tête que tout retard dans cette mise en sécurité, tout retard dans cette prise en charge équivaut à une perte de chance pour chaque enfant concerné. Le groupe CRCE K soutient donc cette proposition de loi, tout en regrettant que la commission en ait affaibli le texte en revenant sur

dans son rapport rendu en novembre dernier,, la Ciivise souligne la difficulté des victimes à être entendues. Seule une victime sur dix révèle les violences au moment des faits, et sur 160 000 enfants victimes de violences sexuelles chaque année, seuls 19 % des cas

et à protéger les victimes, qui, souvent, craignent pour leur sécurité, celle de leurs enfants, voire celle de leurs agresseurs. Il nous faut saluer l’action du législateur et des pouvoirs publics tout en gardant à l’esprit l’ampleur des travaux que nous devons continuer à mener. de ces chantiers. Elle doit en effet évoluer et s’adapter afin de toujours mieux protéger les victimes. Le texte que nous examinons aujourd’hui vise à prolonger cette politique volontariste d’aide et de protection des victimes. Je me réjouis que, sur la quasi totalité des articles,

je ne vois pas de difficulté à ce que la suspension de l’autorité parentale soit effective jusqu’à l’obtention d’un jugement définitif sur les faits incriminés, dès lors qu’un recours auprès du juge aux affaires familiales reste possible pour le parent mis en examen. Je comprends l’inquiétude de notre rapporteure quant à la longueur des procédures pénales, mais le délai maximal de six mois ne me paraît pas pertinent au regard des faits dont le parent est soupçonné d’être l’auteur, et dont la gravité emporte une possible

voilà ce qui nous réunit de nouveau pour l’examen, en deuxième lecture, de la proposition de loi visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales. Ce texte consensuel a été adopté à l’unanimité par l’Assemblée nationale, en première lecture tout d’abord, après avoir fait l’objet d’une réécriture transpartisane réalisée en lien avec le ministère de la justice, et le 13 novembre dernier, lors de son deuxième examen. Les députés ont recherché l’équilibre en reprenant des apports importants du Sénat tels que l’exonération du parent bénéficiaire d’une ordonnance de protection de communiquer tout changement de résidence à l’autre parent, l’interdiction de présenter une demande en rétablissement de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement avant la fin d’un délai de six mois suivant le jugement de retrait devenu irrévocable ou encore l’obligation, pour le juge, de motiver spécialement sa décision en cas de non suspension du droit de visite et d’hébergement d’un enfant dans le cadre d’un contrôle judiciaire prononcé pour violences intrafamiliales. La commission des lois du Sénat, par la voix de sa rapporteure, dont je tiens à souligner le travail de qualité, a quant à elle également fait un pas en direction de nos collègues députés en adoptant quatre articles sans modification. En revanche, et fort malheureusement, subsiste entre nos deux assemblées un point de désaccord majeur, puisqu’il porte sur l’article 1 de la présente proposition de loi, qui élargit aux faits d’agression sexuelle ou de crime commis sur son enfant les principes et les modalités de suspension de l’autorité parentale et de ses attributs en cas de poursuite par le ministère public, de mise en examen par le juge d’instruction ou de condamnation, même non définitive,

Cette suspension provisoire, telle que l’ont souhaitée les députés, serait effective jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, éventuellement saisi par le parent poursuivi, ou jusqu’à la décision de non lieu ou jusqu’à la décision de la juridiction de jugement. La commission a considéré que l’absence de limite dans le temps posait problème au regard de la présomption d’innocence et du droit de chacun de mener une vie normale. Un vote conforme aurait pourtant permis une adoption rapide et définitive de ces dispositions par le Parlement, ce que nous ne pouvons que regretter. Comme le groupe RDPI le recommandait en première lecture, il semble indispensable de sécuriser la situation de l’enfant. Le retour au texte issu de l’Assemblée nationale, qui conditionne le maintien de cette suspension à une décision du juge, nous semble répondre à cet impératif. Nous vous présenterons un amendement dans ce sens,

de ces violences qui leur laissent des séquelles psychologiques et physiques graves. Cette proposition de loi visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales, déposée par notre collègue députée Isabelle Santiago après un travail avec la Chancellerie, nous revient en deuxième lecture, après avoir été à nouveau adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale. Ce texte constitue un pas de plus vers la protection des enfants. Il s’inscrit dans un législatif qui, peu à peu, se consolide. à chaque fois au rendez vous, monsieur le garde des sceaux, nous continuons d’espérer une grande loi sur la protection des femmes et des enfants, ainsi que sur les violences intrafamiliales, comme le soulignait ma collègue Laurence Rossignol en première lecture. La loi du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste a opéré un changement attendu dans l’appréhension pénale des violences sexuelles perpétrées sur des victimes mineures en insérant dans le code pénal de nouvelles infractions d’agressions sexuelles autonomes sur mineurs de moins de 18 ans dans le cas de l’inceste. Rappelons que c’est le groupe socialiste qui avait, par amendement, proposé de relever l’âge du non consentement de 15 à 18 ans dans le cadre du crime d’inceste. Lors de l’examen de cette loi, de nombreuses associations avaient reproché au Parlement de ne pas être allé assez loin, notamment sur la question du retrait de l’autorité parentale, autorité trop souvent instrumentalisée par le parent auteur de crime ou d’inceste afin de garder une emprise sur la ou les victimes. Lors de l’examen de la loi

avait proposé par amendement le retrait de l’autorité parentale, notamment dans le cadre de l’ordonnance de protection. Cette disposition avait alors été rejetée. C’est regrettable, car de nombreux mois ont été perdus.

présentencielle, soit pour un crime commis sur la personne de l’autre parent, soit pour une agression sexuelle incestueuse ou pour un crime commis sur la personne de son enfant, soit enfin

Les dispositions relatives aux violences conjugales sont ainsi supprimées, comme la suspension de l’autorité parentale de plein droit pendant toute la durée de la procédure. Nous le regrettons, et nos regrets sont partagés par d’autres groupes au Sénat, comme nous avons pu l’entendre. Un vote conforme aurait par ailleurs permis d’appliquer le nouveau dispositif plus rapidement.

Nous attendons encore des évolutions en termes de droit de l’enfant, notamment le droit pour celui ci d’être entendu ou d’être automatiquement assisté par un avocat lors de toute procédure judiciaire le concernant. Les annonces gouvernementales du mois de mai dernier, relatives notamment à la création de pôles spécialisés, vont certes dans la bonne direction, mais, au delà des textes, la question des moyens se pose. Il ne faudrait pas, au prétexte que l’argent manque, limiter la portée de cette proposition de loi.

la disposition retenue par la commission des lois et Mme le rapporteur serait elle de nature à porter atteinte aux droits et à la protection de l’enfant ? Elle ne leur porte atteinte en rien. En revanche, elle préserve

en France, entre 10 % et 20 % la proportion d’adultes ayant subi de telles violences lorsqu’ils étaient mineurs : des millions de nos concitoyens sont donc directement concernés.

Mes chers collègues, ce sujet est on ne peut plus sensible. En la matière, nous devons légiférer avec la plus grande prudence en nous en tenant à deux objectifs clairs : préserver l’intérêt supérieur de l’enfant et valoriser la parole des victimes. Ces deux enjeux doivent primer toute autre considération. À ce stade de la navette parlementaire, plusieurs avancées ont été entérinées. Je pense notamment à l’article 2, qui prévoit l’automaticité du retrait de l’autorité parentale et de son exercice, lorsque des violences ou un crime ont été commis contre l’autre parent ou lorsque l’enfant a subi un viol. Sur ce point, la navette a permis d’aboutir à un dispositif à la fois efficace et équilibré. Ce n’est pas encore le cas pour l’article 1. Mme la rapporteure de la commission des lois, dont je tiens à saluer le travail consciencieux et rigoureux, a proposé de rétablir la version adoptée par le Sénat en première lecture, en conservant au juge aux affaires familiales la faculté de se prononcer sur la suspension provisoire de l’autorité parentale. J’entends certains de nos collègues – et ils sont nombreux – insister pour que ce texte soit adopté et promulgué le plus rapidement possible, afin qu’il produise ses effets au plus vite et qu’un maximum d’enfants soient ainsi mis à l’abri.

J’en suis convaincu : mieux vaut prendre le temps nécessaire pour concevoir la meilleure loi possible plutôt que de se hâter et d’adopter un texte probablement moins efficace ou moins équilibré. Certes, l’Assemblée nationale a envoyé un message fort en votant sa version du texte à l’unanimité ; mais l’unanimité d’une chambre ne remet pas en cause le bicamérisme. Le Sénat doit poursuivre son travail de manière

plus, il n’est pas rare que l’enfant victime soit contraint de maintenir des liens avec le parent violent : cela peut paraître absurde et révoltant, mais c’est pourtant le cas. Trop longtemps, l’idée selon laquelle on peut être un mari violent, mais un bon père, a prévalu, jusque dans nos tribunaux. texte entend corriger cela. Bien entendu, nous ne partons pas de rien. Je pense par exemple à la loi du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille, dont vous étiez déjà la rapporteure, chère Marie

Cette proposition de loi, que nous examinons en deuxième lecture, entend renforcer notre arsenal juridique afin de répondre à un enjeu que nous faisons tous nôtre ici : mieux protéger les enfants. Concrètement, le présent texte permettra de suspendre plus facilement et plus rapidement, non seulement l’autorité parentale, mais aussi les droits de visite et d’hébergement. Les faits concernés sont des crimes, parmi les plus graves, qui visent directement l’enfant ou l’autre parent. Ce texte apporte toutefois des limites nécessaires – je pense par exemple à la possibilité, pour le parent concerné, de saisir le juge aux affaires familiales pour réexaminer la décision ce texte prévoit une suspension provisoire en cas de poursuite et un retrait total en cas de condamnation, mais il instaure un cas de délégation forcée de l’exercice de l’autorité parentale à un tiers.

demande est formulée de longue date par toutes les associations de victimes : elle sera bientôt enfin satisfaite. Enfin, je me félicite de l’adoption conforme de l’article 3 , issu d’un amendement que j’avais déposé en première lecture en commission. Cet article pose le principe de la suspension du droit de visite et d’hébergement de l’enfant dans le cadre d’un contrôle judiciaire comprenant une interdiction d’entrer en contact ou d’une obligation de résider hors du domicile du couple.

Je tiens ici à saluer le travail et la recherche de compromis de notre rapporteure, Marie Mercier, dont l’engagement sur ce sujet est connu de tous.

conservés. Dans la rédaction de l’Assemblée nationale, la saisine du juge aux affaires familiales pour réexamen de la mesure de suspension est en effet facultative et prise sur l’initiative du parent concerné ; mais est ce vraiment une mauvaise chose ? L’article 1 n’a vocation à s’appliquer que dans les affaires les plus graves : le parent poursuivi sera forcément assisté d’un avocat, qui saura lui rappeler la nécessité de saisir le juge aux affaires familiales. À ce titre, si

Fernique. Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, en France, un enfant meurt sous les coups de ses parents chaque semaine ; un enfant est victime de violences sexuelles toutes les trois minutes.

On te croit » : c’est ce que chaque victime mérite de ressentir. Mais puisque les violences sont systémiques, croire les victimes n’est qu’une étape de la lutte contre ces violences. Nul n’ignore que des mesures ont déjà été prises. Je salue évidemment les annonces du plan de lutte contre les violences faites aux enfants pour les années 2024 à 2027, présenté en décembre dernier. Mais, si ce plan va dans le bon sens, beaucoup reste à faire, y compris pour faciliter le recueil des témoignages. Il est tout aussi primordial que nous protégions les enfants victimes de violences intrafamiliales. D’une part, cette protection suppose une augmentation de moyens, y compris pour accélérer le traitement des affaires par notre système judiciaire, qui souffre toujours du sous investissement chronique des dernières décennies. D’autre part, nous devons rendre notre législation plus protectrice pour les enfants victimes de violences. La loi de 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes est malheureusement restée muette sur plusieurs aspects ; la proposition de loi de notre collègue députée Isabelle Santiago entend donc aller plus loin, dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Grâce au travail constructif et transpartisan mené en première lecture, le présent texte contient des avancées que les élus du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires soutiennent sans réserve. C’est le cas, par exemple, du retrait total de l’autorité parentale en cas de condamnation pour crime commis sur l’autre parent, agression sexuelle incestueuse ou crime commis sur l’enfant.

confrontation qui se révèle traumatique pour la victime. Ce n’est là qu’un exemple des nombreuses failles que les travaux monumentaux de la Ciivise ont permis d’identifier et qui permettent aux violences de persister à l’abri des regards. Sous la coprésidence de Nathalie Mathieu et d’Édouard Durand, cette commission a relevé un grand nombre d’obstacles persistants, s’opposant à une poursuite pénale efficace. Il apparaît ainsi que la vidéo des premières auditions des victimes reste très peu visionnée par les juges.

je m’adresse donc à vous : qu’allez vous faire pour mettre fin aux manquements identifiés par la Ciivise ? En attendant, nous allons veiller à ce que le présent texte, que nous soutenons pleinement, soit le plus protecteur possible pour les victimes.

ainsi que les apports de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences faites aux enfants, dont nous venons d’entendre les louanges, lesquels ont permis d’enrichir ce texte. Chaque année, 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles, le plus souvent dans le cercle familial, comme l’a rappelé l’ancien président de la Ciivise, le juge des enfants Édouard Durand. Parallèlement, le nombre de plaintes reste beaucoup trop faible pour lutter contre ce système d’impunité intrafamiliale, qui profite toujours aux agresseurs. avons nous perdu tant de temps pour protéger ces enfants, pour les mettre à l’abri de parents destructeurs ? Pourquoi leur statut de victimes a t il été si longtemps ignoré, alors qu’il devait être au centre de nos préoccupations ? Le temps est venu de prendre conscience de la gravité et des conséquences de ces violences sur le développement de l’enfant. Le présent texte va enfin permettre de renforcer la procédure de retrait de l’autorité parentale c’est une mesure de bon sens, qui doit devenir la règle pour les cas de crimes et d’agressions sexuelles. Alors députée, notre collègue Valérie Boyer avait d’ailleurs proposé une mesure identique à l’Assemblée nationale

Nous sommes en 2024 et l’accumulation des textes législatifs a entraîné une inertie insupportable pour les victimes. Tous les jours ou presque, des conjoints violents se servent des enfants. Tous les jours ou presque, ces enfants sont réduits au rang d’objets de transaction, qui permettent aux parents violents de maintenir une tyrannie quotidienne. Ces enfants, qui vivent dans un foyer violent, sont restés trop longtemps invisibles et inaudibles pour les pouvoirs publics et les institutions judiciaires. Pourtant – nous le savons

jamais assez : un parent violent ne peut être considéré comme un bon parent. Une société qui ne sait pas protéger ses enfants est une société malade et la violence faite à ces enfants relève aussi de notre responsabilité en tant que législateur. Je souhaite que ce texte provoque une prise de conscience telle que chacun se sente investi d’une responsabilité face à ces problèmes, bien trop longtemps passés sous silence. Le combat pour la protection des enfants est l’affaire de tous. Je voterai donc cette proposition de loi, qui replace l’enfant au centre du système judiciaire.

fratrie. L’extension de la suspension de l’autorité parentale à toute la fratrie éviterait d’avoir à mener une procédure longue et coûteuse pour protéger chacun des enfants. protégés du même coup. Dans le cas où les autres enfants n’ont pas été victimes de crime de la part du parent accusé, la protection de l’ensemble de la fratrie permettrait d’éviter que le parent maltraitant ne maintienne son emprise sur les autres enfants ou ne réitère sur eux ses agissements passés

au parent poursuivi de saisir le JAF. Les désaccords manifestes entre nos deux chambres et dans notre hémicycle le prouvent : il n’est pas évident de trouver un équilibre entre la protection de l’enfant et le droit de mener une vie familiale normale.

Les parents représentent 86 % des auteurs présumés de maltraitance et 160 000 enfants sont victimes chaque année de violences sexuelles. Qu’allons nous dire à toutes ces victimes ? Qu’au regard de la présomption d’innocence, il était disproportionné de les maintenir éloignés de leurs parents violents ?

des parents à l’égard de l’autre parent en présence de l’enfant. En 2020, huit femmes victimes de violences sur dix avaient des enfants. En 2021, douze enfants ont été tués dans un contexte de violences conjugales

de l’autorité parentale dès le stade des poursuites, pour les agressions sexuelles incestueuses, les crimes commis contre l’enfant et les crimes commis contre l’autre parent, ce jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, saisi par le parent poursuivi, la décision de non lieu du juge d’instruction ou la décision de la juridiction de jugement. Nous parlons d’un sujet majeur et ce mécanisme nous semble aller pleinement dans l’intérêt de la protection de l’enfant. Nous ne saurions faire preuve de

sur la nécessité de permettre la suspension de l’autorité parentale du parent inculpé pour des violences sexuelles incestueuses ou pour un crime commis sur la personne de l’autre parent. Mais, comme en première lecture, la majorité sénatoriale souhaite toujours limiter

cette suspension serait levée. Le parent poursuivi pour violences graves retrouverait alors le plein exercice de tous les droits dont il disposait auparavant. Il se peut qu’il soit condamné peu après : ses droits lui seraient de nouveau retirés, toujours dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Mais pendant quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois, ce dernier risque de se retrouver dans une situation et d’être exposé à des violences. C’est précisément le type de situation que nous devons éviter. Pour protéger l’enfant de potentielles violences, il faut permettre une suspension provisoire au delà de six mois, comme l’ont prévu nos collègues députés. De plus, il faut suspendre provisoirement l’exercice de l’autorité parentale du parent condamné pour des violences majeures sur l’autre parent en attendant la décision définitive. Cette mesure a elle aussi été adoptée à deux reprises, à l’unanimité, par l’Assemblée nationale.

telle mesure ne suffit pas à ériger la protection des enfants en priorité absolue. Elle signifie qu’au bout de six mois un enfant victime d’inceste ne serait plus protégé

de la Ciivise : la suspension de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi pour viol ou agression sexuelle incestueuse sur la personne la protection des enfants doit nous guider ; le bien être supérieur de l’enfant doit être notre boussole. Un Français sur dix a été victime d’inceste durant son enfance, soit plus de 5 millions de femmes et d’hommes. Les chiffres et les statistiques font écho au quotidien et au passé traumatique de millions de Français et Françaises. Les enfants victimes ne sont pas les seuls concernés par ce dispositif : les frères et sœurs d’une même fratrie seraient également protégés, et ce jusqu’à la décision du juge. La suspension de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement s’appliquera nécessairement à tous les enfants sur lesquels

n 4 rectifié et 12 rectifié sont des amendements de repli qui tendent à ne rétablir que le mécanisme de suspension en cas de crime et d’agression sexuelle incestueuse. La commission a réaffirmé son attachement au fait qu’un juge aux affaires familiales soit systématiquement saisi pour prolonger

Comme vous y allez ! Je le dis de façon très claire : il n’est aucunement question que l’on puisse inverser la charge de la preuve ! Je sais que c’est une revendication de plus en

vous proposez, par ces multiples amendements, de rétablir la version de l’article 1 adoptée par l’Assemblée nationale, qui crée deux mécanismes

Il s’appliquerait jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, saisi dans un délai de six mois à compter de la décision pénale. Je vous rejoins évidemment sur la nécessité de prévoir que le mécanisme de suspension de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale s’applique aux crimes et aux agressions sexuelles incestueuses dont peut être victime un enfant. C’est d’ailleurs une demande de la Ciivise, et le Gouvernement y voit un moyen efficace pour protéger les enfants d’un parent potentiellement violent ou abuseur dans l’attente de la décision

Par ailleurs, vous souhaitez supprimer l’obligation pour le procureur de saisir le juge aux affaires familiales, afin qu’il statue sur cette suspension automatique de l’exercice de l’autorité parentale. Ce point fait débat entre les deux assemblées

dans des délais qui ne sont pas ceux que vous avez indiqués – le juge aux affaires familiales pour demander à être rétabli dans ses droits.

lorsque l’enfant a assisté aux faits. Il s’appliquerait jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, saisi dans un délai de six mois à compter de la décision pénale.

un enfant meurt sous les coups de ses parents tous les cinq jours et 160 000 enfants sont victimes chaque année de violences ou d’inceste.

portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir en France, mes collègues Daniel Fargeot, Hervé Marseille et Franck Menonville ont été enregistrés comme ne prenant pas

Évelyne Renaud Garabedian, Bruno Rojouan et Jean Pierre Vogel souhaitaient voter pour. Acte est donné de vos mises au point, mes chères collègues. Elles figureront dans l’analyse politique du scrutin concerné. L’ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée,

Madame la présidente, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, la politique de protection des consommateurs exige la mise en œuvre de moyens permettant de rechercher et de sanctionner les pratiques ne respectant pas leurs droits.

depuis 2016, les associations d’usagers du système de santé agréées ont la possibilité d’intenter des actions de groupe pour les dommages causés par des produits de santé. même année, l’action de groupe s’applique aussi à la lutte contre les discriminations, à la protection des données personnelles et aux dommages environnementaux. En 2018, l’action de groupe en matière de consommation a également été étendue aux litiges relatifs à la location de biens immobiliers. Le panorama actuel de l’action de groupe en droit français est donc complexe : il repose sur une diversité de régimes dont les règles procédurales, les préjudices indemnisables et les modalités de réparation ne sont pas uniformes. En outre, le bilan des actions de groupe reste décevant. En effet, seules trente deux actions ont été intentées depuis 2014, et aucune d’entre elles n’est allée jusqu’au bout de la procédure, qui, pour rappel, est divisée en deux phases : le jugement sur la responsabilité, dans un premier temps, puis l’indemnisation des membres du groupe, Plusieurs des actions introduites n’ont pas prospéré pour des raisons de recevabilité ; quelques unes ont débouché sur des accords transactionnels. Les causes de cette situation ont été bien analysées par les députés Laurence Vichnievsky et Philippe Gosselin dans le rapport qui fut à l’origine de la présente proposition de loi ; je veux saluer leur implication sur ce sujet. L’action de groupe est un outil qui doit permettre de faciliter l’accès des justiciables à la justice. Au regard de cet objectif, le Gouvernement partage le constat des auteurs de ce texte quant à la nécessité de lever les obstacles aux actions de groupe, qui sont essentiellement liés à leur complexité.

Ce texte prévoit notamment une unification des différents régimes d’action de groupe ; un champ matériel désormais universel, quels que soient les intérêts en vertu desquels l’action est exercée une qualité pour agir très largement ouverte ; la désignation de juridictions spécialisées appelées à connaître des actions de groupe ; la création d’une amende civile pour faute dolosive ayant causé des dommages sériels ; la suppression de l’obligation de mise en demeure

plusieurs modifications importantes ont été apportées. Je pense en particulier à la limitation de la reconnaissance de la qualité pour agir aux seules associations agréées, à la suppression de l’amende civile, à la généralisation d’une mise en demeure obligatoire préalable ainsi qu’à l’application de la loi aux seules actions dont le fait générateur est postérieur à sa publication. Plusieurs de ces évolutions répondent aux préoccupations du Gouvernement ; je remercie le rapporteur d’en avoir tenu compte dans le cadre de ses travaux. Je pense notamment au risque de sanctions

que les entités qui se lancent dans une action de groupe auront les moyens de la poursuivre tout au long de la procédure – qui peut être longue.

d’une mise en demeure préalable à toute introduction d’une action de groupe, le Gouvernement est plus réservé, compte tenu du risque associé d’allongement des procédures, sans bénéfice évident. ne paraît pas adaptée aux actions en cessation introduites à l’encontre de pratiques illicites particulièrement préjudiciables aux intérêts des consommateurs ou à leur santé. Pour ce qui est de l’application de la loi aux seuls faits générateurs postérieurs à sa publication, cette restriction a pour conséquence d’exclure les situations en cours et de priver les victimes des dommages concernés de cette voie de réparation que constitue l’action de groupe.

inhérent au nouveau régime de l’action de groupe. Le Gouvernement s’en remettra donc à la sagesse du Sénat… Proverbiale ! … pour ce qui est de trouver un point d’équilibre garantissant les intérêts des victimes sans fragiliser les acteurs économiques.

À cet égard, le Gouvernement se félicite que le texte issu des travaux de la commission emporte, sur l’initiative de son rapporteur, une transposition complète et conforme de la directive. loi exige des associations habilitées qu’elles mettent en place des mesures d’information et de publicité ; elle instaure un contrôle des conflits d’intérêts par

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, garantir aux justiciables une voie de protection efficace de leurs intérêts, tout en préservant les opérateurs économiques d’un risque réputationnel potentiellement dévastateur pour leur activité : tel est le délicat chemin de crête qu’arpente le législateur depuis la création, voilà une décennie, de l’action de groupe. Le débat sur l’opportunité de son introduction est bien plus ancien ; on peut le dater d’il y a au moins quarante ans… Malgré son âge, ses termes n’ont pas beaucoup évolué : d’un côté, la protection des droits des justiciables, notamment des consommateurs, implique la mise à leur disposition de voies de droit efficaces leur permettant d’obtenir réparation de préjudices, y compris quand ceux ci sont d’un faible montant de l’autre, notre système judiciaire, auquel incombe la protection de l’activité des opérateurs économiques contre d’éventuelles actions malveillantes visant uniquement à les déstabiliser, nécessite que l’action de groupe « à la française » ne soit pas calquée sur la américaine et sur ses dérives. Ce cadre étant posé, la proposition de loi déposée et rapportée par nos collègues députés Laurence Vichnievsky et Philippe Gosselin se caractérise, à rebours de l’équilibre délicat recherché par le législateur il y a une décennie de cela, par une certaine forme de radicalité assumée.

Il serait déraisonnable d’affirmer que l’action de groupe constitue aujourd’hui une voie procédurale plébiscitée, mais je veux souligner que la prémisse d’un échec de l’action de groupe me paraît contestable. actions de groupe ont été engagées depuis 2014, et l’inégale qualité des demandes a eu pour effet qu’un certain nombre d’entre elles ont été déclarées irrecevables par le juge. Pour autant, ce bilan mitigé peut en partie être attribué à la nécessaire phase d’appropriation qu’implique la création d’une telle procédure. Par ailleurs, certaines actions de groupe ont prospéré et permis l’indemnisation d’un préjudice, parfois dans le cadre d’un accord amiable. Ne partageant manifestement pas cet avis, les auteurs – et rapporteurs pour l’Assemblée nationale – de la proposition de loi ont souhaité encourager le recours aux actions de groupe.

de la qualité pour agir, enfin, celle ci étant très largement ouverte, y compris à des associations représentant un nombre limité de personnes. Dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, la position d’équilibre jusqu’à présent recherchée par le législateur semblait donc reléguée aux oubliettes au profit d’une proposition de loi nettement plus radicale, trait renforcé par l’introduction d’une amende civile en cas de faute intentionnelle ayant causé un ou plusieurs dommages à plusieurs personnes physiques ou morales placées dans une situation similaire. Face à un dispositif qu’elle a jugé quelque peu déséquilibré, la commission s’est en conséquence attachée à retrouver le chemin de crête qui a, jusqu’alors, guidé les pas du législateur. Les amendements qu’elle a adoptés ont ainsi visé trois objectifs. Premier objectif : resserrer un cadre juridique excessivement lâche. Ainsi, tout en acceptant l’universalisation des préjudices indemnisables, mais également, dans son principe, celle

par des acteurs ne disposant que de peu de moyens de défense. À cet égard, le fait que le droit de la responsabilité ne soit pas modifié est sans importance, puisque le risque qu’emporte l’introduction d’une action de groupe porte non pas tant sur l’engagement indu de la responsabilité que sur le coût procédural et réputationnel qu’une telle action publique ne manque pas d’entraîner. Surtout, la commission a significativement resserré les conditions d’octroi de la qualité pour agir. Au régime juridique très libéral résultant des travaux de l’Assemblée nationale, qui permettrait à un grand nombre d’acteurs, y compris malveillants, d’agir dans de nombreux domaines, la commission oppose

L’instauration d’un agrément nous a ainsi paru incontournable pour garantir le sérieux et la transparence des personnes ayant qualité pour agir, notamment en matière de prévention des conflits d’intérêts notre dispositif est peut être perfectible, mais il me semble largement préférable à une simple attestation sur l’honneur, qui n’a d’autre valeur que celle de l’encre utilisée pour la rédiger. Deuxième objectif : prévenir les risques juridiques que soulève le dispositif. Le premier d’entre eux concerne naturellement l’amende civile prévue à l’article 2 , dont le Conseil d’État a justement relevé les difficultés constitutionnelles qu’elle pose.

un problème de méthode : l’insertion, presque par effraction, d’une mesure qui modifie très significativement le droit de la responsabilité civile dans un texte de procédure, sans étude d’impact préalable, paraît extrêmement problématique.

Au bénéfice de ces quelques aménagements, la commission a adopté un texte qui présente l’immense avantage – trop rare de nos jours ! – de simplifier effectivement le droit. Elle n’a néanmoins pas souhaité faire dévier le législateur du chemin de crête qu’il s’est employé à arpenter jusqu’à présent. a été modifié par la commission, le texte qui est aujourd’hui soumis à votre examen, mes chers collègues, vise donc à préserver et à garantir un juste équilibre entre la protection des droits des justiciables et la sécurité juridique des opérateurs économiques. utile pour permettre à l’action de groupe, dont la vocation n’est pas d’être un épiphénomène juridique ni une procédure banalisée, de trouver sa voie. La parole

la consécration de l’action de groupe en droit français a été tardive. Son refus a d’ailleurs été plus souvent dogmatique que juridique. Il s’est tout d’abord agi d’un refus de principe : on lui opposait l’adage suivant lequel « nul ne plaide par procureur ».

S’il fallait encore nous en convaincre, le droit comparé suffirait en un rien de temps à montrer que certains dogmes n’ont pas fait illusion dans l’esprit du législateur étranger : je pense au modèle américain bien sûr, mais aussi à ceux du Québec, de l’Argentine, du Brésil, du Portugal, de l’Angleterre, ou encore de l’Espagne et de la Suède.

il est impératif, d’une part, d’éviter toute forme de marchandisation de l’action judiciaire et, d’autre part, de contenir un accroissement excessif du risque judiciaire pour les entreprises.

à dire de conjurer l’une des dérives observables du modèle américain. Ce constat justifie également que les associations ayant qualité pour engager une action doivent répondre à certains critères. Nous suivrons donc la position du rapporteur, qui n’a souhaité ouvrir ce mode de recours qu’à des associations soumises à un agrément. Reste la question de l’amende civile, disposition que proposaient nos collègues députés et que notre commission a souhaité ne pas conserver. Nous comprenons évidemment le sens et l’opportunité de ce dispositif, s’agissant de sanctionner l’auteur d’un dommage lorsqu’il a délibérément commis une faute en vue d’obtenir un gain ou une économie et lorsque la réparation du préjudice ne suffit pas à neutraliser le profit qu’il a réalisé. Sur ce point, nous aurions tendance à suivre l’avis émis tant

Pour conclure mon propos, je souhaite évoquer une dernière difficulté qui a trait à l’application de la future loi. Nous avons été alertés par de nombreux professionnels au sujet de l’article 3, qui restreindrait le nouveau régime de l’action de groupe aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité ou le manquement

comme cela a été rappelé, l’action de groupe, qui a pour objectif de faciliter l’accès au droit des victimes d’un même dommage n’ayant pas toujours la possibilité d’agir seules en justice dans des contentieux souvent techniques,

L’action de groupe a ensuite été étendue, en 2016, aux litiges en matière de santé, d’environnement, de protection des données personnelles et de discrimination au travail, puis, en 2018, aux litiges relatifs à la location d’un logement.

Les très fortes contraintes juridiques qui entourent cette procédure dans notre pays semblent avoir eu pour conséquence d’empêcher toute action de groupe, ou presque, de prospérer. Aussi, sans tomber dans les dérives que peuvent connaître les États Unis, il est proposé, par ce texte, de créer un régime juridique unifié des actions de groupe

à la cessation d’un manquement ou à la réparation d’un préjudice subi à raison dudit manquement. Il s’agit par ailleurs d’indemniser tous les préjudices, qu’ils soient corporels, matériels ou moraux, d’ouvrir la qualité pour agir et de maintenir la possibilité de recourir à la médiation pour faciliter l’indemnisation des victimes et favoriser le désengorgement des tribunaux.

les dispositions figurant dans la directive du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives, qui visent à protéger les intérêts collectifs des consommateurs

ferait courir aux opérateurs économiques. La commission a également supprimé l’amende civile, au sujet de laquelle le Conseil d’État avait émis de fortes réserves. Malgré des modifications substantielles, notre groupe considère que l’économie du texte est préservée. Dix années après la création de la procédure de l’action de groupe, nous serons vigilants pour que la version issue de nos débats permette une utilisation efficace de ce droit par les justiciables français. C’est la raison pour laquelle nous voterons cette proposition de loi.

ministre de l’économie sociale et solidaire, le Parlement votait le projet de loi portant création de l’action de groupe à la française. L’objectif de ce dispositif était double : permettre aux victimes de se rassembler pour parler d’une seule et même voix ; permettre aux victimes de faire reconnaître le préjudice subi et de faire valoir leur droit à réparation. La volonté du législateur était de rééquilibrer une relation contractuelle trop défavorable aux consommateurs. Cette ambition était plus que louable. Elle était même noble. Pourtant, dix ans après, force est de constater que cette avancée législative n’a, hélas ! pas eu les effets escomptés. Le législateur de 2014 avait souhaité limiter le champ de l’action de groupe au domaine de la consommation, et ce principalement parce qu’il voulait éviter les écueils et dérives manifestes ayant émergé dans le cadre des en droit anglo saxon. Par la suite, le régime de l’action de groupe a lentement évolué la loi du 18 novembre 2016 l’a étendu aux discriminations au travail, aux questions environnementales et au respect des données personnelles. Puis, en 2018, son champ a été ouvert aux préjudices causés par la location d’un logement. Pourtant, malgré ces extensions successives, l’action de groupe est restée peu usitée. Depuis sa création, cela a été rappelé, ce droit n’a été activé qu’une trentaine de fois seulement. Six procédures ont débouché sur un résultat positif dans trois d’entre elles, le défendeur a été déclaré responsable, tandis qu’un accord amiable a pu être trouvé dans les trois autres. Six procédures qui prospèrent et aboutissent en dix ans, c’est peu C’est même trop peu, alors que, dans la même période, nous avons assisté à l’essor exponentiel de la vente par correspondance et des transactions commerciales sur internet, singulièrement pendant la crise sanitaire du covid Afin de dresser un bilan des premiers pas de l’action de groupe au sein de notre législation, les députés Philippe Gosselin et Laurence Vichnievsky ont rendu, le 11 juin 2020, un rapport exhaustif et précis. Selon nos collègues députés, le caractère relatif du succès des actions de groupe serait dû à de multiples freins. Tout d’abord, notre droit en la matière serait trop complexe, puisque le régime en question n’a pas été unifié. Ensuite, son champ d’application serait trop restreint. Enfin, le faible nombre d’associations habilitées à agir – une quinzaine seulement – n’aurait pas été de nature à favoriser le recours à ce dispositif.

C’est sur la base de la transcription juridique de ces propositions que Philippe Gosselin et Laurence Vichnievsky ont déposé le 15 décembre 2022 la proposition de loi que nous examinons aujourd’hui. Cette initiative parlementaire a ensuite été largement enrichie en première lecture à l’Assemblée nationale. le texte est passé à quarante et un articles dans la version qui a été transmise au Sénat. Cette version, mes chers collègues, était pleinement de nature à nous satisfaire. D’abord, elle simplifiait le droit existant en l’assouplissant. elle créait une action de groupe au régime universel. En outre, elle permettait l’élargissement de la qualité à agir, du champ d’application et du préjudice indemnisable. Elle instaurait par ailleurs une sanction civile en cas de faute intentionnelle de l’entreprise ayant causé des dommages sériels à plusieurs individus. Enfin, elle ouvrait la voie à la spécialisation de tribunaux judiciaires en matière d’action de groupe, choix que nous voyons plutôt d’un bon œil, mais qui nécessitera une vigilance certaine, afin que les juridictions en question soient justement réparties sur le territoire national. Les associations de consommateurs avaient salué ce texte transpartisan, et la Défenseure des droits, Claire Hédon, s’était réjouie de sa qualité. Le soutien unanime de la société civile et des différents groupes politiques de l’Assemblée nationale n’a cependant pas pleinement convaincu notre rapporteur, que notre rapporteur, que je remercie néanmoins pour la qualité de son travail et pour les nombreuses auditions qu’il a bien voulu organiser. En effet, lors de nos travaux en commission, il a fait le choix de réduire substantiellement la portée de cette proposition de loi en rigidifiant la procédure de recours aux actions de groupe, tout en restreignant largement la capacité des associations à agir en la matière. Il a par ailleurs choisi de supprimer la sanction civile réprimant les fautes intentionnelles ayant engendré des dommages sériels, et borné dans le temps l’application de cette loi aux seuls nouveaux litiges,

qui plaçaient de grands espoirs dans nos travaux. L’expertise d’usage de ces associations aurait pu – aurait dû – nous convaincre toutes et tous de la pertinence de la philosophie du texte issu de l’Assemblée nationale.

au risque de laisser perdurer les insuffisances de la législation actuelle. L’objectif affiché de cette proposition de loi était de rééquilibrer le rapport de force entre ce que l’on appelle familièrement le pot de terre et le pot de fer. À cet égard, le texte issu de la commission des lois du Sénat semble beaucoup moins ambitieux que nous ne l’aurions souhaité. Je tiens à rappeler un élément essentiel une entreprise qui respecte la loi, le droit et tout lien contractuel qu’elle aurait pu nouer n’a absolument rien à craindre d’un élargissement du champ de l’action de groupe. Très juste ! Seuls les opérateurs qui se savent délibérément en tort ou potentiellement fautifs

Si notre législation se fait suffisamment dissuasive et si elle pousse mécaniquement les acteurs économiques à se conduire de manière vertueuse, ne devrions nous pas nous en féliciter ? Notre souci principal ne devrait il pas se trouver dans la défense du consommateur, et dans la capacité de la victime à faire valoir ses droits ? Pour répondre à ces questions et atteindre ces objectifs, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain a déposé quatre amendements. Ceux ci visent principalement à revenir à une rédaction plus volontariste et à une approche plus inclusive et plus ambitieuse de cette proposition de loi, dans la droite ligne du travail produit par nos collègues de l’Assemblée nationale. Nous avons fait le choix de concentrer principalement nos efforts sur l’habilitation des associations à agir en matière d’action de groupe, ainsi que sur l’application de la présente proposition de loi aux litiges intentés antérieurement à son entrée en vigueur. Si nous n’avons pas réussi à convaincre notre collègue rapporteur au stade de l’examen du texte en commission des lois, nous formons le vœu que les débats de ce jour nous permettent de converger pour en revenir à la philosophie et à la mouture du texte issu des travaux de l’Assemblée nationale. C’est à l’aune de l’accueil qui sera réservé à nos amendements et à ceux qui ont pour objet de revenir à l’esprit initial de la proposition de loi que les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain décideront de leur vote. Mes chers collègues, nos travaux ont suscité de l’espoir chez nombre de justiciables et de consommateurs spoliés. Certains vous ont même peut être écrit pour vous le signifier. Nous avons aujourd’hui l’occasion d’offrir aux Françaises et aux Français

Est ce vraiment le droit qui nous empêche aujourd’hui de mettre en œuvre des actions de groupe ? Ceux qui ont lu le rapport du Conseil d’État – ils sont quelques uns dans cet hémicycle – ont pu y lire qu’au Portugal les actions de groupe, bien qu’étant largement admissibles,

Voilà bientôt dix ans qu’elle est entrée dans notre droit, et avec elle l’ambition de faire de chaque citoyen un procureur privé. Pour autant, elle n’est pas devenue un réflexe naturel en France,

par le fait que cette action – il faut bien le reconnaître – ne s’inscrit pas dans notre tradition juridique : en France, l’intérêt général est défendu par l’action publique, par le procureur, par l’État, et non par des actions privées. Ensuite, l’exemple du système américain a fait craindre, chez nous, la multiplication de procédures dilatoires hostiles, mettant à mal les entreprises. Tout cela est vrai. Pourtant, l’action de groupe à la française, telle que nous la concevons, a du sens. Elle représente la création réussie d’un équilibre entre l’accès des justiciables à la justice, d’une part, et la protection des défendeurs contre les actions malveillantes,

de groupe, régime juridique en constante évolution, a perdu sa cohérence ; il était temps de la lui rendre. Ainsi la proposition de loi que nous examinons

Bien que technique, cette proposition de loi traite d’un sujet fondamental pour l’évolution de notre société. Les améliorations qu’elle apporte nous paraissent décisives. Aussi le groupe Les Indépendants votera t il en faveur de son adoption.

souvent nous entendons dire que nous adoptons trop de lois, compliquant toujours davantage la vie des Français. Ne parle t on pas d’une passion normative française ? Seulement, contrairement à ce que l’on pense, cette triste habitude ne remonte pas à des temps récents : Alexis de Tocqueville, au XIX siècle, s’en plaignait déjà. Aussi, je tiens à saluer le travail mené à l’Assemblée nationale par nos collègues Laurence Vichnievsky et Philippe Gosselin, qui ont voulu simplifier les règles régissant les actions de groupe afin de rendre cette procédure plus accessible à nos concitoyens.

ainsi été estimé que, pour la seule année 2022, 141 recours collectifs y ont été résolus pour un montant de 4,77 milliards de dollars. Ces chiffres sont à comparer aux trente deux ou trente cinq actions de groupe engagées en France depuis 2014. Peu importe cette différence comptable, ce qui en ressort, c’est un bilan plus que décevant.

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, « les enfants exposés au valproate présentent un risque élevé de troubles graves du développement et du comportement ». Cette phrase, on peut la lire sur les notices des médicaments qui contiennent du valproate, substance active d’un médicament antiépileptique. Et l’alerte est plus que fondée,

la Dépakine a été prise en cours de grossesse. Conséquence : des milliers d’enfants sont nés avec des malformations de leur colonne vertébrale, de leur crâne, de leur cœur. D’autres présentent des symptômes d’autisme ou des troubles d’hyperactivité.

Pourtant, elle est susceptible d’améliorer la protection des citoyennes et des citoyens, qui sont trop souvent impuissants face à un acteur dominant comme l’est une grande entreprise. Comme l’illustre tristement le scandale de la Dépakine, un enfant né avec des malformations peut difficilement traduire un grand laboratoire pharmaceutique en justice. La victime ne dispose guère d’informations sur l’étendue du problème, tandis que l’entreprise peut mobiliser d’importantes ressources pour se défendre. En permettant aux victimes d’être représentées par un acteur tiers, l’action de groupe améliore l’accès à la justice. Mais

C’est pourquoi nous soutenons, bien évidemment, l’initiative de nos collègues députés Laurence Vichnievsky et Philippe Gosselin, qui vise à faciliter le recours aux actions de groupe.

lieu, ils ont souhaité rendre la procédure plus équitable et plus efficace, par exemple en instituant des tribunaux judiciaires spécialisés en matière d’action de groupe. Le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires souscrit pleinement à ces propositions, qui ont été améliorées grâce à l’important travail transpartisan mené au Palais Bourbon. Afin de lutter contre l’asymétrie entre les grandes entreprises, d’une part, et les citoyennes et citoyens, de l’autre, nous avons déposé une série d’amendements pour aller plus loin

libre aux États membres d’aller plus loin ! C’est le choix qu’ont fait d’autres pays. Au Portugal, le droit d’introduire une action de groupe est même inscrit dans la Constitution. que de vous cacher derrière un tel argument, mes chers collègues, assumez ce que vous tentez de faire : créer des obstacles aux actions de groupe afin de protéger les intérêts des grandes entreprises Vous vous opposez ainsi à toute amélioration de la situation actuelle, dans laquelle la victime de mauvaises pratiques d’une grande entreprise n’a que peu de chances d’obtenir réparation.

Je vous remercie

les « garde fous » visant à éviter « les dérives constatées dans d’autres pays », aux « graves conséquences pour les entreprises » – je cite toujours Pierre Moscovici –, ont dévitalisé cette promesse d’une justice accessible au plus grand nombre.

la première action de groupe à avoir passé l’étape de la première instance sera peut être la première réelle déception engendrée par une procédure trop complexe depuis ses premiers jours. Mme Véronique Legrand, maître de conférences à l’université de Caen, nous a rappelé quels freins procéduraux

Où est donc passée la souplesse censée être au fondement de cette procédure qui devait, disait on, satisfaire l’impératif d’accessibilité de la justice ? Le désir de justice s’éloigne, et les brèches sont béantes quand le justiciable, même organisé, s’en prend à plus fort que lui, lorsqu’il s’agit d’une multinationale.

soit, comme l’explique M. Cédric Musso, directeur de l’action politique de l’UFC Que Choisir, « le périmètre de la loi a été, une interprétation restrictive, considérablement réduit

Se pose alors la question de savoir si les pouvoirs publics ont conscience que ce texte en demi teinte affaiblit la place de Paris au bénéfice d’autres capitales européennes qui jouent le jeu d’instaurer une “vraie” [action de groupe]

est vidé de son sens par le risque d’octroi de dommages et intérêts punitifs. Nous sommes loin du compte ! En effet, la présente proposition de loi ne remet pas en cause certains vices de la loi Hamon

chers au cœur des Percherons –, ce qui offre à leurs pays un avantage compétitif indéniable pour attirer vers eux tous les demandeurs d’une action représentative. Le projet de loi manque là une occasion de hisser la place judiciaire française au premier rang des dispositifs européens d’action collective ; c’est vraiment dommage. Les affaires

M. Daniel Salmon. Depuis le début de la discussion, nous avons beaucoup entendu dire que cette proposition de loi permettait d’élargir les actions de groupe à tous les domaines

qui ne concerne en réalité qu’une partie des situations où des centaines – voire des milliers – de personnes se trouvent lésées à cause d’un manquement d’une entreprise. Prenons l’exemple du Mediator, ou celui des organismes de certification de prothèses mammaires. Dans ces Dans ces affaires, il n’y a pas eu de manquement à des obligations légales ou contractuelles, mais les entreprises ont manqué à leur devoir de vigilance. De même, si Total a été condamné dans l’affaire du naufrage du pétrolier, ce n’est pas parce que l’entreprise avait directement manqué à une obligation légale ou contractuelle, mais parce qu’elle avait manqué de contrôler l’état du navire qui transportait du pétrole pour son compte avant de s’échouer, causant une catastrophe environnementale que tous les Bretons ont subie. Ce n’est pas pour rien que le code civil dispose que toute personne ayant commis une faute doit réparer le dommage qui en résulte. La jurisprudence a reconnu qu’un manquement au devoir général de prudence ou de vigilance constitue également une telle faute. Au civil, le devoir de réparation n’est donc pas conditionné à la violation d’une quelconque disposition légale ou contractuelle, et pour cause.

on irait à rebours de la position de la commission, ce qui me paraît poser des difficultés certaines. L’élargissement proposé est déjà considérable ; il convient donc de procéder avec prudence, afin de ne pas soumettre des opérateurs économiques à un risque réputationnel qui serait indu.

pour objet d’élargir le champ d’application de l’action de groupe aux manquements au devoir général de prudence ou de vigilance. À À l’évidence, un tel élargissement n’est pas adapté à ce type de recours, comme cela a d’ailleurs été parfaitement expliqué par M. le rapporteur, compte tenu notamment de la difficulté à qualifier ce type de manquements, qui de surcroît s’apprécient dans de très nombreux cas au regard de situations particulières – j’en prends pour exemple le devoir de vigilance du banquier.

Telle est la question que je me suis posée quand la majorité sénatoriale, en commission, a fait adopter cet article, qui a justement pour objet de protéger les entreprises de poursuites dans certains cas.

C’est ce que regrette d’ailleurs la CFDT, qui note notamment que les actions de groupe seraient plus efficaces en la matière que des actions sérielles devant les conseils de prud’hommes. Les actions de groupe en ces matières ne sont pas craintes par les organisations syndicales ; bien au contraire, elles sont très demandées. vient d’être condamné, voilà à peine deux semaines, pour le fonctionnement défectueux des conseils de prud’hommes, où les délais de jugement sont bien trop longs. Plutôt que de craindre que les actions de groupe en matière de droit du travail privent les prud’hommes de leurs compétences, nous devons veiller à ce que tout le monde ait un accès effectif à la justice,

Celui qui limite le champ des actions de groupe à la lutte contre les discriminations ou celui qui ouvre la possibilité d’agir collectivement en matière de protection des données personnelles et pour obtenir la cessation d’un manquement et la réparation de tout dommage causé à des personnes sous l’autorité d’un employeur

Premièrement, en matière de santé, nous avons été alertés quant au très grand risque que pourraient encourir des professionnels de santé disposant de faibles moyens de défense face à des actions de groupe destinées à salir leur réputation. Entendons nous bien, mes chers collègues :

de l’amendement n° 26, pourraient toujours faire l’objet d’actions de groupe. En revanche, nous estimons que le risque réputationnel que pourraient en particulier encourir des professionnels de santé justifie d’exclure ceux ci du champ de l’action de groupe et d’en rester au champ actuel. Je souhaite ailleurs répondre à l’argument parfois avancé consistant à affirmer que, le « fond du droit » de la responsabilité n’étant pas modifié par la proposition de loi, ces changements procéduraux seraient sans effet sur l’engagement de la responsabilité des professionnels de santé. C’est exact, mais c’est oublier que le véritable coût d’une action de groupe est réputationnel : quel patient irait consulter un médecin dont le nom figure injustement au registre des actions de groupe, dont je rappelle qu’il est créé par la présente proposition de loi ? Dans le cas où la responsabilité du professionnel en question ne serait pas reconnue, comment compenser le préjudice ainsi subi ? L’action de groupe « à la française » ne nous paraît pas devoir s’orienter vers ce type de dérives. Deuxièmement, en matière de droit du travail, il nous a semblé qu’une ouverture indiscriminée de l’action de groupe risquerait en particulier de dessaisir les conseils de prud’hommes de pans non négligeables du contentieux, ce qui serait un effet de bord particulièrement fâcheux de cette réforme, les prud’hommes rendant la justice au plus près des intérêts des salariés et des employeurs. Il nous a également semblé,

si le champ de l’action de groupe était étendu, on pourrait voir de telles procédures intentées devant le juge pour des dommages occasionnés par la pratique de professionnels résultant de conditions d’organisation du service

Nous commençons, avec cet article, l’examen des conditions requises pour avoir qualité pour agir. En d’autres termes, cet article répond à la question suivante : « qui peut introduire une action de groupe ? » Or cette définition est primordiale pour faciliter le recours aux actions de groupe et, par ricochet, l’accès à la justice.

Élargir la qualité pour agir est primordial si l’on veut améliorer l’accès à la justice des citoyennes et des citoyens. En aucun cas nous ne devrions conditionner la qualité pour agir à l’obtention d’un quelconque agrément. La perte par

Enfin, dans un État de droit, l’élargissement de la qualité pour agir ne devrait représenter aucun problème. L’introduction d’une action de groupe ne saurait en elle même causer de préjudice aux entreprises mises en cause, car la présomption d’innocence vaut aussi pour cette procédure

Pour aider les associations à introduire des actions de groupe, ce qui relève de l’intérêt général, la Défenseure des droits a d’ailleurs proposé de créer un fonds spécifique. Malgré tout, leurs capacités resteraient limitées.

Afin de limiter le nombre de tels cas, il est donc important d’ouvrir plus largement la qualité pour agir. Plus il y a d’associations pouvant introduire une action de groupe, moins il y aura de personnes lésées privées d’un accès praticable à la justice. Pour faire court, élargir la qualité pour agir permet d’améliorer l’accès à la justice. La

seules les associations agréées et les organisations syndicales représentatives auraient la faculté de déposer une demande d’action de groupe. les associations déclarées depuis deux ans au moins, dont l’objet est la défense d’intérêts spécifiques, sont constituées aux seules fins de rassembler la force de plusieurs plaignants ; aussi les associations agissant pour au moins cinquante personnes ou cinq collectivités territoriales. Comprimer la liste des organisations pouvant intenter de telles procédures revient à annihiler les bénéfices de l’élargissement des matières auxquelles

Croyez vous que nos concitoyens engageraient de telles procédures par simple malveillance, comme si réclamer réparation n’était pas long, fastidieux et coûteux ? On ne se présente pas devant le juge par plaisir ! Il faut sortir de cette logique

En outre, concernant les cas de discrimination à l’égard des candidats, cet amendement vise justement à ouvrir les actions de groupe aux associations régulièrement déclarées depuis deux ans, contre cinq ans actuellement.

Le contentieux une action de groupe est possible, depuis peu, en matière de données personnelles : il y a là une réelle avancée. Il faut maintenant aller plus loin. Les travailleurs des plateformes subissant des préjudices similaires ou de même nature doivent pouvoir se coaliser face aux plateformes numériques qui rivalisent d’ingéniosité pour les priver de leurs droits.

La fraude et l’évasion fiscales pénalisent certes les finances publiques et rompent le pacte social, c’est une évidence, mais la fraude fiscale et boursière mine aussi le pacte social dans les entreprises en éludant une partie de la richesse créée ou en sacrifiant l’outil productif à quelques actionnaires au profit d’une valorisation boursière rehaussée.

qui sont en première ligne pour créer de la valeur doivent être en première ligne pour en tirer profit. Le profit n’est pas réservé aux actionnaires ! Il doit, sinon ruisseler, du moins bénéficier aux travailleurs des augmentations de salaires convenables. Ouvrir les actions de groupe aux syndicats représentatifs d’une entreprise

à Mme Nathalie Goulet. Il s’agit d’étendre la possibilité de l’action de groupe aux organisations syndicales à vocation générale d’exploitation agricole et aux organisations des pêcheurs et des professions de la mer.

Vous vous méfiez des collectivités territoriales se regroupant en associations afin de faire valoir leurs droits ; dont acte. Mais pour quelle raison entretiendriez vous une telle défiance pour cinq collectivités qui engageraient une procédure par l’entremise d’un avocat ?

Quand bien même reconnaître la qualité à agir d’un avocat dans le cadre de l’action de groupe lui conférerait la qualité de demandeur au sens de la proposition de loi, il agirait dans l’intérêt des personnes physiques ou morales qui l’auraient mandaté pour ce faire. L’article 411 du code de procédure civile ne dit pas autre chose : « Le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure.

représentant des intérêts soit d’au moins cinquante personnes physiques, soit d’au moins cinq personnes morales de droit privé inscrites au registre du commerce et des sociétés depuis au moins deux ans, soit d’au moins cinq collectivités territoriales ou groupement de collectivités.

de la qualité pour agir tel que défini à l’Assemblée nationale paraît excessivement large. La commission s’est précisément attachée à restaurer un agrément permettant de garantir le sérieux et de contrôler la transparence des associations qui engageront des actions de groupe. Cette garantie est fondamentale afin d’éviter que des associations créées en peu de temps

Vous préféreriez donc des associations constituées le matin même, qui comptent cinq adhérents et auxquelles on demande une attestation sur l’honneur griffonnée sur un bout de papier, dont la seule valeur est celle de l’encre qui a

Quelle audace, en effet ! Cet amendement tend à inclure les syndicats agricoles et les syndicats de pêcheurs

qu’un manquement est commis par toute personne agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de son activité professionnelle, il pourrait faire l’objet d’une action de groupe,

effet de créer une situation de conflit d’intérêts. Comment le juge pourra t il déterminer si le financement a pour objet ou pour effet d’influencer l’action de groupe ?

demande une déclaration d’intérêts complexifierait inutilement l’engagement d’une action de groupe. Elle porte intrinsèquement en elle les risques de susciter du contentieux en cas d’allégation de faux, de reporter la charge de la preuve d’un éventuel conflit d’intérêts sur le défendeur et d’allonger la procédure en mêlant les voies civiles et les voies pénales. Par ailleurs, elle n’est pas de nature à contribuer à un véritable

J’y suis défavorable, pour plusieurs raisons. Il s’agit d’une condition inutile, car la régularité de la situation fiscale ne conditionne aucunement le bien fondé de l’action. En outre, les dérives des actions de groupe que vous évoquez ne sont pas liées à la situation fiscale du demandeur. Par ailleurs, cette obligation serait source d’insécurité juridique, puisque la sanction de son non respect n’est pas précisée. En tout état de cause, il n’apparaît pas pertinent de conditionner la recevabilité d’une action à la régularité de la situation fiscale du demandeur. Enfin, le juge a toujours la possibilité d’enjoindre aux parties de communiquer telle ou telle pièce s’il l’estime nécessaire.

AA afin de préciser le rôle et les pouvoirs du juge dans le contrôle de l’absence réelle de conflit d’intérêts en tant que condition de recevabilité de l’action de groupe. Cette réécriture s’inscrit dans la continuité des travaux de votre commission, qui a renforcé le texte en prévoyant un contrôle par le juge du conflit d’intérêts. Il s’agit simplement de veiller à ce que ces dispositions soient pleinement opérationnelles en précisant la procédure, afin d’éviter la naissance de contentieux inutiles. L’amendement tend à préciser que le contrôle de l’absence de conflit d’intérêts sera effectué par le juge saisi d’une demande en ce sens. Le juge pourra solliciter la production de toutes pièces permettant de vérifier cette absence. Le contrôle par le juge sera ainsi pleinement effectif, et la directive pleinement transposée.

de groupe, adopté à l’unanimité, contenait la recommandation n° 10 suivante : « Supprimer l’obligation de mise en demeure préalable pour les actions de groupe en matière d’environnement, de protection des données personnelles et de discrimination.

Si la mise en demeure a effectivement pour effet de rallonger la procédure de l’action de groupe, elle peut néanmoins permettre d’éviter certaines procédures indues. » Monsieur le rapporteur, chers collègues de la majorité sénatoriale, qu’est ce qu’une « procédure indue » ? Pourquoi craindrait on ceux qui réclament justice ?

oblige les victimes présumées à avertir l’entité qu’elles entendent attaquer et à attendre de quatre à six mois, selon les matières, avant de saisir la justice. Pendant ce temps, le préjudice demeure et la situation pourrit.

y lit : « Ce délai rallonge considérablement la durée des procédures alors que le manquement à une obligation légale ou contractuelle pourra continuer à porter préjudice pendant la durée de la procédure.

J’espère donc que les sénatrices et sénateurs du groupe Les Républicains reviendront sur leur position pour suivre les préconisations du rapport d’information coécrit par un député… des Républicains. Par ailleurs, l’obligation que vous prévoyez aurait pour conséquence que la procédure serait plus lourde qu’elle ne l’est actuellement. En effet, la mise en demeure n’est pas obligatoire pour les actions de groupe en matière de santé ou pour les contentieux locatifs

Saint Antoine et Les Avirons, l’eau du robinet était impropre à la consommation. L’agence régionale de santé y avait trouvé, entre autres, des bactéries fécales. Pour éviter de boire de l’eau contaminée, les citoyennes et les citoyens n’avaient d’autre solution que d’acheter de l’eau en bouteille telle situation ne pouvait pas durer. Pour autant, le distributeur d’eau n’a rien entrepris pour mettre rapidement un terme à cette contamination. C’est pourquoi une association de défense des consommatrices et consommateurs a décidé d’engager une action de groupe.

cela soit évidemment primordial pour éviter des dommages supplémentaires, l’organisation du système judiciaire ne le permet pas toujours. Et le sous investissement chronique des dernières années n’aide pas, bien sûr, car il allonge encore davantage les délais.

il paraît préférable de laisser aux juges une marge d’appréciation suffisante dans l’appréciation du délai raisonnable dans lequel il peut être procédé à la cessation du manquement. Pour ces deux raisons, je demande le retrait

la procédure à suivre dans la phase de jugement sur la responsabilité, en rapprochant les dispositions de la présente proposition de loi du droit en vigueur. D’une part, le droit en vigueur dispose que, en cas

précipitée du jugement sur la responsabilité et complexifier la procédure. D’autre part, le même article 1 prévoit que le délai d’adhésion des personnes dont les intérêts ont été lésés au groupe susceptible de recevoir une indemnisation

Cet amendement vise à faire en sorte que le jugement statuant sur la responsabilité puisse faire l’objet d’une publicité une fois qu’il a acquis un caractère définitif, c’est à dire qu’il ne peut plus faire l’objet d’un appel ou d’un pourvoi en cassation.

statuant sur la responsabilité. Néanmoins, je ne suis pas favorable à la réduction du délai maximal de publicité de cinq ans à deux ans. En effet, certains préjudices nécessitent, du fait de leur nature même, un délai d’adhésion plus long que deux ans : c’est le cas, par exemple, en matière de préjudices

Ce pouvoir d’instruction permettrait de réduire le déséquilibre informationnel qui existe systématiquement entre l’entreprise mise en cause et les personnes lésées. En effet, la première dispose nécessairement de plus d’informations, par exemple sur les risques d’un procédé industriel, et il appartient à la partie demanderesse de démontrer que l’entreprise n’a pas correctement évalué les risques, donc qu’elle a manqué à prévenir un dommage. Afin de l’aider dans cette démarche, les juges pourraient, par exemple, demander la remise de certains documents. Dans d’autres pays, les pouvoirs des juges en la matière vont beaucoup plus loin que ce qui est prévu par nos procédures civiles et pénales.

Cela signifie qu’actuellement, lorsqu’une action de groupe est intentée, un juge de la mise en état est désigné. Ce juge a le pouvoir d’ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction qu’il juge utile, conformément aux dispositions des articles 789 et